ministre de l'économie et des finances.

je suis très heureux de vous présenter le projet de loi de finances pour 2020, dans un contexte économique marqué par des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine et un ralentissement prononcé de la croissance mondiale, aussi bien aux États-Unis et en Chine qu'au niveau européen.

ai redit à quel point nous étions opposés aux sanctions infligées aux viticulteurs français. Il faut que ces derniers sachent qu'ils peuvent compter sur le soutien du gouvernement français, et sur mon soutien,

Nous sommes également confrontés à un ralentissement de la croissance européenne. De ce point de vue, je rappelle que la France tire son épingle du jeu : elle fait mieux que les autres pays européens, puisqu'elle maintient un niveau de croissance élevé, un niveau d'investissement important et une attractivité qui est désormais la meilleure de tous les pays membres de la zone euro. Le dernier point général sur lequel je veux insister, après avoir évoqué les tensions commerciales et le ralentissement de la croissance dans la zone euro, est la persistance de taux d'intérêt faibles, voire négatifs,

Dans ce contexte général de ralentissement de la croissance mondiale et de taux d'intérêt bas, voire négatifs, quelle est la politique que nous vous proposons à travers le projet de loi de finances pour 2020 ? C'est une politique d'innovation, une politique pour le travail et une politique de poursuite du rétablissement de nos finances publiques. Face au ralentissement de la croissance, la seule politique qui nous paraît valable est celle de l'investissement dans l'avenir et de la poursuite d'une politique de l'offre, qui, je le redis, a commencé à donner des résultats, avec la création d'un demi-million d'emplois dans notre pays, la restauration de marges de manoeuvre industrielles et le maintien d'une croissance solide. Nous avons donc maintenu des choix fiscaux en faveur des entreprises. Il y aura 1 milliard d'euros de baisse nette d'impôts sur les entreprises en 2020. L'intégralité des allégements de charges, quel que soit le niveau de salaire, seront maintenus, sachant que ces allégements ont été renforcés au 1 octobre dernier, puisqu'il n'y a plus aucune cotisation patronale au niveau du SMIC.

La visibilité sera maintenue, puisque le cap des 25 % de taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises sera atteint en 2022, comme le Président de la République s'y était engagé. Les entreprises dont les chiffres d'affaires sont les plus modestes verront leur impôt sur les sociétés baisser plus rapidement en 2020 que les autres, mais toutes les entreprises, quel que soit le niveau de leur chiffre d'affaires, bénéficieront bien d'une baisse de l'impôt sur les sociétés dès 2020, selon une trajectoire qui les amènera au en 2022. Autre baisse d'impôt pour les entreprises : le prélèvement sur les entreprises affecté au financement des chambres de commerce et d'industrie diminuera. Nous nous y étions engagés, et nous tiendrons cet engagement. Je veux également profiter de cette intervention pour rassurer les chambres de commerce et d'industrie : elles ont fait un travail très important pour se moderniser et s'engager dans une transformation en profondeur. J'ai toujours indiqué que nous vérifierions que la trajectoire prévue est supportable pour les chambres ; nous organiserons bien un point d'étape en 2020 pour nous assurer que toutes les chambres de commerce et d'industrie arrivent à supporter cette transformation. Je rappelle enfin que la suppression du prélèvement « France Télécom » permettra de rendre près de 30 millions d'euros aux chambres pour accompagner la transformation de leur modèle.

40 milliards d'euros de baisses d'impôt au total. Nous sortons de la période de matraquage fiscal qu'ont connue les entreprises et les ménages, en France, depuis plusieurs années.

C'est pour cette raison que nous avons décidé de sanctuariser le crédit d'impôt recherche, auquel nous ne toucherons pas. Nous avons simplement pris en compte les remarques de la Cour des comptes sur le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement,

Cette politique d'innovation est aussi ce qui nous a conduits à céder un certain nombre d'actifs que l'État détenait dans des entreprises, en particulier La Française des jeux, dont je viens, ce matin, de lancer la cotation. La La privatisation de La Française des jeux est un immense succès : un succès populaire- plus d'un demi-million de Français y ont participé -, un succès pour La Française des jeux, qui a montré sa solidité, un succès pour la place financière de Paris, qui a montré qu'elle était attractive. C'est bien la preuve qu'il est possible de réconcilier les Français avec l'investissement dans les entreprises, qu'il est possible de permettre à une entreprise de se développer dans de bonnes conditions sur le marché tout en conservant

laisser les entreprises commerciales se développer, leur donner les moyens d'un tel développement, tout en gardant un droit de contrôle de l'État, et concentrer l'effort de l'État sur ce qui est vital pour les générations à venir, l'innovation et l'investissement dans l'intelligence artificielle, dans les énergies renouvelables, dans le stockage des données, dans tout ce qui fera, demain, la souveraineté de notre pays. Notre deuxième grande orientation est celle de la rémunération du travail.

vous proposons également de voter, dans ce budget, des baisses d'impôt en matière de taxe d'habitation, qui s'ajoutent à notre politique de meilleure rémunération du travail. S'il y a une leçon à retenir de la crise des « gilets jaunes », c'est qu'une immense majorité de Français aspirent à la dignité par le travail, à la juste rémunération de leur activité ; ils veulent pouvoir vivre bien du travail qu'ils font et du salaire qu'ils touchent. Toutes les mesures que nous avons prises depuis près de trois ans s'inscrivent exactement dans cette orientation : la revalorisation de la prime d'activité, 100 euros de plus par mois au niveau du SMIC pour tous ceux qui travaillent,

C'est une question de justice, de reconnaissance du travail et d'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Récompenser le travail, c'est aussi avoir la lucidité de voir à quel point, dans certains services publics- je pense aux hôpitaux -, les économies qui ont été demandées depuis des années ont pu provoquer des difficultés, des blocages, voire des souffrances de certains personnels. Le plan pour l'hôpital public qui a été annoncé par le Premier ministre, d'une ampleur inédite, vise précisément à mieux récompenser le travail de ce personnel hospitalier auquel nous devons tant. Des primes seront donc versées pour soutenir le personnel hospitalier : 100 euros nets par mois dès 2020 pour les aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées, 800 euros nets de prime annuelle pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et dans sa proche banlieue, 300 euros de prime annuelle distribués directement par les hôpitaux. Nous avons également accepté, avec le ministre des comptes publics, de reprendre une partie de la dette des hôpitaux, ce qui va permettre de dégager des moyens supplémentaires pour que les hôpitaux publics puissent, soit assainir leur situation financière, soit investir dans des travaux du quotidien indispensables

la première hausse interviendra non pas au 1 janvier 2020, mais au 1 juillet 2020, de façon à laisser aux professionnels le temps de s'adapter. Ceux-ci auront droit, en outre, à un certain nombre de compensations que nous mettrons en oeuvre

Toutes ces compensations répondent à des semaines de discussions avec les professionnels concernés par la suppression de cet avantage fiscal. Deuxième niche que nous réduirons le mécénat d'entreprise. Grave erreur ! Nous voulons l'encadrer. Nous avons donc baissé le taux de défiscalisation de 60 % à 40 % pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros, ce qui ne concerne, je le rappelle, que 78 grandes entreprises.

Le troisième dispositif que nous modifions est l'avantage lié à la déduction forfaitaire spécifique. Cet avantage sera plafonné, ce qui permettra de réaliser une économie de 400 millions d'euros dès 2020. Ce plafonnement est proposé dans le cadre Voilà les économies de dépense publique que nous faisons ! Cependant, je constate que, chaque fois que nous mettons en oeuvre de telles économies, tous ceux qui les réclament par ailleurs votent contre, ce que je trouve regrettable. Le sens des responsabilités devrait les conduire à voter les réductions de dépense publique qui financent les baisses d'impôt qu'attendent tous les Français ! Le troisième point est logique vu ce que je viens de dire : c'est le rétablissement de nos finances publiques. Nous avons engagé, avec Gérald Darmanin, depuis trois ans, le rétablissement des finances publiques françaises.

! Il n'y a pas que les chiffres ! Ces chiffres montrent que nous rétablissons nos finances publiques : nous stabilisons la dette et nous baissons le déficit public. Certains diront, à juste titre, que nous le faisons à un rythme qui est plus lent que ce qui était prévu. C'est vrai je pense qu'il est raisonnable d'adapter le rythme du rétablissement des finances publiques tant à la conjoncture internationale qu'à la situation sociale du pays. Nous ne perdons pas le fil de notre politique, qui vise à rétablir les finances publiques françaises. Nous rétablirons les finances publiques françaises ! Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une crise sociale majeure dans notre pays. On ne peut pas faire comme si des millions de Français n'avaient pas réclamé une amélioration de leurs conditions de vie. Et on ne peut pas faire comme si n'existait pas la crise internationale qui a mené à un ralentissement profond de la croissance mondiale, aux États-Unis comme dans la zone euro

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs,

à notre conviction en matière de maîtrise des dépenses publiques et à la transformation structurelle de nos politiques publiques, qui nous ont permis de réduire à la fois nos impôts et nos déficits. Les résultats sont là ; ils sont incontestables.

L'ampleur inédite de la réponse que nous avons apportée à l'urgence économique et sociale nous conduit sans doute à faire des modifications, mais sans changer de cap. Je voudrais d'ailleurs souligner la sincérité avec laquelle nous présentons désormais les comptes de la Nation- cette sincérité est saluée

que présente le Gouvernement à la représentation nationale. Cela fait deux fois, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement ne présente pas de décret d'avance,

dans la République française, n'avait jamais supprimé un impôt de 22 milliards d'euros ; c'est ce qu'aura fait le Président de la République ! Il s'agit d'une réforme historique, vous le savez, et j'imagine que nous prendrons le temps, au Sénat, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale, d'en discuter,

par l'accélération de la transition écologique. Les crédits alloués à la transition écologique et aux transports augmenteront de 3 milliards d'euros sur le quinquennat et de 800 millions d'euros dès 2020, et la trajectoire prévue par la loi d'orientation des mobilités

lorsque le Sénat souhaitera l'examiner, dans le PLFSS, mais il comportera bien une exonération fiscale en plus de l'exonération de cotisations sociales. L'allocation aux adultes handicapés sera revalorisée de 1,3 milliard d'euros sur le quinquennat

la TVA pour la France. Nous savons tous que la fraude est un coup de poignard au pacte républicain. Nous travaillerons sur la liste des États non coopératifs en cas d'évasion fiscale. Nous proposerons une disposition très intéressante sur la domiciliation fiscale des dirigeants, qui entraînera sans doute un certain nombre de

diminue le déficit, réduit les impôts, garantit la croissance, lutte contre la fraude fiscale, simplifie la vie des Français, réforme la fiscalité locale.

d'orientation des finances publiques. Le scénario de remontée des taux d'intérêt est significativement revu à la baisse par rapport au programme de stabilité d'avril, dont nous avions souligné le caractère conservateur.

avec une amélioration de 3 milliards d'euros permise par une hausse spontanée des recettes qui permet de « couvrir » une augmentation de 7,7 milliards d'euros de la norme de dépenses pilotables et des investissements d'avenir

Actuellement oui, au regard des marchés, mais en cas de retournement de conjoncture ? Les dépenses des ministères dépassent tous les objectifs fixés précédemment. Vous affirmez que les dépenses sont inférieures à ce qui était prévu en loi de finances initiale

! Lors de l'examen de la loi de programmation des finances publiques, Gérald Darmanin avait affirmé des ambitions auxquelles nous pouvions souscrire. Elles sont aujourd'hui abandonnées. Le ministre

après un long temps de travail en commission. Je veux souligner, en préambule, l'implication de mes collègues de la commission des finances, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux, qui, depuis plusieurs semaines, étudient en détail les mesures budgétaires et fiscales de ce projet de loi de finances pour forger leurs convictions. Ils ont ainsi entendu 488 personnes au cours de plus de deux cents heures d'audition, la commission y consacrant plus de quarante heures de réunions plénières. Les commissions saisies pour avis ont également conduit des auditions diverses, en particulier ministérielles. Tout ce travail préparatoire sera particulièrement utile pour éclairer nos débats, dans le respect du délai constitutionnel contraint de vingt jours.

elle ne serait plus que de 1,4 % en 2019 et de 1,3 % l'an prochain. De plus, les incertitudes tant internationales qu'européennes, avec la perspective du choc lié au Brexit- sans parler des risques internes liés à d'éventuels conflits sociaux, comme notre pays a pu en connaître avec la crise des « gilets jaunes » et comme il s'en profile encore -, pèsent incontestablement sur cette prévision de croissance. Elles devraient nous inciter à la prudence, tant un retournement de conjoncture exposerait nos finances publiques. Or, de la prudence, ce projet de loi de finances en manque considérablement. Il ne laisse aucune marge de manoeuvre en cas d'évolution négative du contexte économique national, européen ou mondial. Comme je l'ai déjà souligné, le Gouvernement s'écarte de la loi de programmation des finances publiques qu'il avait fait adopter à l'automne 2017 et choisit de ne pas la réviser pour ne pas souligner l'ampleur de ses renoncements et son manque d'ambition pour nos finances publiques. Malgré des taux d'intérêt très bas, qui allègent considérablement la charge de la dette- elle devrait diminuer de 3 milliards d'euros en deux ans -, l'endettement public frôlera les 100 % du produit intérieur brut en 2020, à rebours de la réduction qui avait été annoncée. budget de renoncement, puisque l'objectif de retour à l'équilibre de nos comptes publics pour la fin du quinquennat est définitivement abandonné. Nous ne respectons pas non plus le minimum de redressement demandé par nos partenaires européens. L'effort structurel est réduit à néant, le Président de la République estimant d'ailleurs que la règle des 3 % du PIB pour notre déficit public relève d'« un débat d'un autre siècle », sans toutefois indiquer quel est son objectif dans ce domaine. Paradoxalement, la France appelle son principal partenaire européen, l'Allemagne, à renoncer à ses objectifs d'équilibre budgétaire, sans s'engager sur ses propres efforts de redressement et sans témoigner de son sérieux budgétaire. Le Gouvernement, qui se targuait, à l'été 2017, d'engager un mouvement sans précédent de baisse de la dépense publique et de réduire les effectifs de l'État de 50 000 postes a dû finalement se confronter à la dure réalité et aux contraintes de l'exercice. Nos concitoyens demandent un véritable socle de services publics, de présence de l'État dans les territoires et de solidarité nationale. Après un budget pour 2019 présenté comme le « budget du pouvoir d'achat », dont on a vu qu'il correspondait bien mal à cet le budget pour 2020 est surtout celui du renoncement et du en matière de déséquilibres ! Le Gouvernement a en effet dû renoncer à nombre de baisses de dépenses qu'il avait envisagées. Pour autant, les dépenses sur lesquelles il choisit d'agir concernent d'abord les politiques sociales, notamment les contrats aidés, le logement social et les aides au logement, ou encore- pour sortir du strict champ de l'État -l'assurance chômage. Seules des manifestations d'ampleur l'amènent à répondre aux demandes sociales au cas par cas, de manière brouillonne et improvisée, comme on a pu le constater avec l'annonce, hier même, d'un prétendu plan Hôpital. Aucune vision d'ensemble n'est en fait proposée. Dans le même temps, s'il ne parvient pas à tenir les objectifs de maîtrise de la dépense qu'il avait lui-même fixés, le Gouvernement n'a pas renoncé à baisser les impôts, mais il en alourdissant le déficit budgétaire ou en espérant des recettes budgétaires des procédures de privatisation d'entreprises publiques- Aéroports de Paris ou Française des jeux -qui, demain, ne produiront donc plus de dividendes pour l'État. On privilégie des intérêts de court terme au détriment des intérêts de long terme de la Nation. Les baisses d'impôts ont visé par priorité les entreprises et les ménages les plus aisés, sans que l'on puisse estimer l'impact de ces mesures, pourtant coûteuses, sur l'activité économique et l'emploi. J'ai conduit, avec le rapporteur général, une étude sur la réforme de la fiscalité du capital, dont il ressort que rien ne permet de mesurer le fameux « ruissellement » qui devait découler de la suppression de l'impôt de solidarité Au total, les contribuables les plus fortunés auront nettement profité de ces réformes sans rien donner en retour. Même en prenant en compte les mesures post-« gilets jaunes », une étude de l'Institut des politiques publiques sur l'effet cumulé des budgets 2018-2020 montre qu'il n'y a eu aucun gain, ou presque, pour les 20 % les plus pauvres, mais qu'il y a eu une hausse de 4 % des revenus disponibles pour le premier centile des contribuables les plus riches. Ce mardi, l'Insee vient de faire paraître une note qui confirme cette analyse. Je proposerai de revenir sur ces réformes néfastes, sans rétablir tel quel le système fiscal antérieur, mais en le modernisant pour qu'il réponde à l'objectif d'équité fiscale auquel nos concitoyens sont très attachés. Tous les contribuables, y compris les plus aisés, doivent participer à la solidarité nationale. La suppression de la taxe d'habitation, qui concernera, à terme, tous les ménages, ne changera pas la situation pour les redevables les plus modestes, qui en étaient, pour bon nombre d'entre eux, exonérés. Selon les données fournies par le ministère de l'économie et des finances lui-même, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés représentera par ailleurs, à elle seule 44,6 % du coût de la réforme, qui s'élève à 17,6 milliards d'euros ! En revanche, cette réforme non financée risque de mettre en péril les recettes de nos collectivités territoriales, qui demandent des garanties sur la pérennité de leurs ressources et une réelle étude de l'impact de ces mesures. Nous en reparlerons lors de la discussion de l'article 5.

à le souligner, pour ne pas dire à le dénoncer, et les dernières péripéties concernant la fiscalité des biocarburants, le Gouvernement n'a pas établi de ligne claire sur ce point. Nous espérons que les débats sur la première partie du PLF seront l'occasion de le faire et, de façon plus générale, de rapprocher nos dispositifs fiscaux du double objectif d'équité sociale et d'utilité dans l'action publique que toute loi de finances se doit, me semble-t-il, de poursuivre. Nous

Alors que notre pays a connu une année de mouvements sociaux inédits, le Gouvernement n'en tient nullement compte dans son projet de loi de finances. S'il entend les revendications populaires qui s'expriment à travers le pays, ce n'est que pour mieux les dévoyer Alors que les associations féministes demandent un budget de 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences que les femmes subissent et pour assurer une réelle égalité, la majorité discute autour d'un Grenelle à faible portée tout en réduisant les crédits du programme « Égalité entre les femmes et les hommes Tandis que les étudiants alertent sur leurs conditions de vie exécrables, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche va baisser pour la première fois depuis 2008, ... Ce n'est pas vrai ! ... alors même que le nombre d'étudiants augmente. Alors que les « gilets jaunes » ont fait part de leur ras-le-bol à l'égard d'une fiscalité injuste pour des services publics qui s'amoindrissent comme peau de chagrin, le Gouvernement répond par un jeu de dupes, en pensant calmer la colère sociale. Si le projet de loi de finances prévoit une baisse de l'impôt sur le revenu, payé par seulement 50 % de nos concitoyens, la TVA, qui est l'impôt le plus injuste et représente pourtant 50 % des recettes du budget de l'État, ne bouge pas. Pour qui la fin du mois commence bien trop souvent le 15, ces 20 % de taxes, ce sont autant de repas qui leur sont retirés de la bouche, autant de jours passés dans le froid, faute de pouvoir payer les factures. À cette détresse que le Gouvernement semble ignorer, aucune réponse n'est apportée

! Pourtant, le tissu associatif joue un rôle crucial pour nombre de nos jeunes, en leur offrant soutien scolaire, accès au sport ou à la culture. Il a permis l'émergence de nombreux sportifs et artistes. Si le Président était attentif aux banlieues, au-delà des deux secondes d'émotion suscitées par le visionnage d'un film, il aurait trouvé chez un artiste comme Kerry James une référence utile pour résumer sa politique : « Incapables de voir loin, on veut pas le bien, quitte à détruire l'intérêt commun. » Et quel manque de vision à long terme ! Les prétendues baisses d'impôts en faveur des plus modestes que le Gouvernement que le Gouvernement concède seront en réalité financées grâce aux taux d'intérêt négatifs auxquels l'État emprunte, qui lui permettent de récupérer 1,6 milliard d'euros. Ce que le Gouvernement donne aujourd'hui, il le reprendra donc demain pour financer la hausse de la charge de la dette. Alors qu'ont surgi sur le devant de la scène la pauvreté et les difficultés dans nos campagnes ainsi que dans les zones périurbaines, le Gouvernement n'en tient nullement compte. Les prix de l'énergie continuent d'augmenter et les petites lignes de trains de fermer ; 200 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté Lorsque la misère n'est pas sublimée par l'art, elle reste invisible aux yeux du Gouvernement. Que c'est beau ! Je n'aborderai même pas la question écologique, tant l'absence d'ambition est criante au vu des enjeux et de l'urgence. Face à ces politiques de casse des solidarités, d'affranchissement des riches de l'effort commun et de pressurage des classes populaires, nos villes et nos départements sont devenus les derniers remparts contre l'épanouissement d'un libéralisme destructeur.

devenaient de simples guichets de l'État, qu'en serait-il des centres de santé, des bibliothèques, du logement social, des équipements sportifs et culturels, en bref de tout ce qui fait la vie au quotidien Le progrès social et humain, ce n'est pas le projet de ce gouvernement. Son projet, c'est la transformation libérale de l'État à tous les échelons, y compris locaux, et notamment municipal. Après la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux communes,

la suppression de la taxe d'habitation opère une nouvelle mise au pas des collectivités. Cette taxe permettait pourtant de développer des politiques de solidarité. Elle offrait aux municipalités la possibilité de mettre en place des politiques redistributives grâce à un impôt progressif

Faire croire que l'on peut leur accorder un cadeau fiscal de cette ampleur sans que cela emporte de conséquences, c'est déjà fort ; faire croire que c'est une mesure de justice sociale, ça l'est encore plus ! Discrètement mais sûrement, l'exonération de la taxe d'habitation a été étendue aux 20 % des ménages les plus riches. Ainsi, 45 % du coût total de la suppression de la taxe d'habitation profitera à ces 6,3 millions de foyers qui n'en ont pas besoin, tandis que les 16 % de foyers les plus modestes, qui ne payent déjà pas la taxe d'habitation, risquent d'être les plus touchés par la casse des services publics consécutive à cette réforme. En effet, l'État devra trouver des budgets à amputer pour compenser sa participation à la réforme de la fiscalité locale.

une destruction de l'État social au profit d'un État réduit à un simple lieu d'administration des affaires du CAC 40, le tout piloté par des hauts fonctionnaires passant du privé au public, et vice versa. Le dernier acte de ce jeu de dupes interviendra- comme par hasard

Par de basses tactiques politiciennes, le Gouvernement esquive le débat et tente d'imposer ses choix. Notre démocratie mérite mieux que cela. Nous ne pouvons pas discuter d'un projet de loi qui opère des choix de société aussi lourds sans jamais réellement les aborder. Les miettes lâchées tantôt aux étudiantes et aux étudiants, tantôt aux personnels hospitaliers, tout en tentant de les diviser, confirment l'extrême fragilité d'un gouvernement qui demeure minoritaire, acculé par la contestation sociale, et qui tente d'imposer ses choix à l'ensemble de la société.

Les amendements que nous proposerons permettront de vérifier qui veut davantage de justice fiscale et sociale, qui veut lutter contre l'accroissement de la richesse des plus aisés

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

16, 16 , 17, 18, 19, 20, 28, 28 , 32 et 33. Les autres articles seraient examinés dans l'ordre normal du dérouleur. Ces demandes de priorité et de réserve seront formulées demain après-midi à l'ouverture de la séance. Elles concerneront également les amendements portant articles additionnels liés aux articles

la taxe d'habitation, je suis bien conscient que mon intervention ne servira à rien, ... Mais non ! ... dès lors que la haute administration, sûre de sa supériorité et figée dans ses certitudes, n'écoutera rien ! Alors on s'en va ! Je le sais, l'affaire est entendue, il paraît qu'il s'agit de tenir un engagement de campagne. Je me permets juste d'alerter une nouvelle fois sur l'absurdité de la suppression de la taxe d'habitation, une absurdité qui coûtera cher à l'État, donc aux contribuables, et qui portera atteinte à l'autonomie des collectivités C'est encore un cadeau fait à ceux qui paient une taxe d'habitation élevée ! Il aurait mieux valu prévoir un allégement forfaitaire pour tous les contribuables. La suppression de la taxe d'habitation coûtera 20 milliards d'euros chaque année.

aucun maire ne pourra calmer les ardeurs dépensières de ceux qui n'auront plus à financer la satisfaction de leurs demandes par le paiement de l'impôt. Bien sûr, il restera les impôts fonciers, mais ceux-ci ne concernent pas tout ne concernent pas tout le monde. La spécialisation de l'impôt dans les collectivités locales, c'est l'injustice garantie ! Vous n'avez pas réussi à supprimer les communes. Aussi avez-vous inventé une arme de destruction massive beaucoup plus dangereuse : la déresponsabilisation. L'État est impécunieux, il ne profite pas des taux bas pour investir des dépenses structurelles à même de favoriser la relance ou de résoudre les différents problèmes de notre société.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà maintenant plus de deux mois que le Gouvernement fait assaut de communication pour vendre à l'opinion publique ce budget comme étant la réponse à la crise des « gilets jaunes

ni même parfois considérés comme faisant partie de la population par un pouvoir jugé technocratique et arrogant, donnant l'impression de prendre des décisions davantage en suivant une logique de « tableau Excel » qu'en étant immergé dans la vie réelle. Ces sentiments sont largement partagés par ceux dont le président Macron a dit un jour qu'ils « ne sont rien » ou qui ne figurent pas parmi les bienheureux « premiers de cordée ». Plus que jamais, notre société est profondément fracturée. la France d'en haut et la France d'en bas » de notre ancien collègue Jean-Pierre Raffarin, la « fracture sociale » pointée en son temps par le candidat Jacques Chirac. La « France périphérique » d'aujourd'hui se révolte et dit sa colère de ne pouvoir mener une vie décente, une vie tout simplement normale. Notre République va mal parce que notre société connaît des inégalités de plus en plus fortes. Les rapports successifs, notre vécu quotidien le démontrent régulièrement. Votre politique, quoi que vous puissiez en dire, aggrave cette situation. En 2018, le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 % pour atteindre 14,7 % de la population ; près d'une personne sur sept vit sous le seuil de pauvreté dans notre pays, la sixième puissance économique mondiale, la troisième sur le plan de l'Union européenne. Concrètement, au-delà de ce pourcentage, ce sont 400 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté, laquelle concerne aujourd'hui plus de 9 millions de nos concitoyens. Ce chiffre en hausse se trouve être le plus élevé depuis 2011 et n'a été dépassé qu'à deux reprises depuis vingt-trois ans, en 1996 et en 2011. Du côté des « premiers de cordée », où en sommes-nous en cette année 2019 ? 2019 ? Ne soyez pas inquiets, mes chers collègues, soyez même enthousiastes, car de ce côté-là tout va bien, merci pour eux ! Ces « premiers de cordée » ont toutes les raisons de se féliciter des choix économiques et fiscaux du gouvernement de M. Macron. Les mesures socio-fiscales mises en place par le Gouvernement en 2018 ont augmenté le niveau de vie des Français de 1,1 %, mais elles ont surtout avantagé les 10 % les plus aisés Cette catégorie a gagné 790 euros de pouvoir d'achat par an en moyenne, contre 130 à 230 euros pour le reste de la population. Les plus grands bénéficiaires des réformes de l'exécutif ont bien sûr été les détenteurs de capital.

Concrètement, cela concerne les foyers fiscaux dont le revenu annuel est supérieur à 700 000 euros. Telle est la réalité, la traduction concrète de vos choix, messieurs les ministres. Après le « grand débat », plus rien ne devait être comme avant. Nous allions entrer dans l'acte II du quinquennat, et ce budget allait donc traduire en mesures concrètes le virage social annoncé. Vous nous dites vouloir rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le récit est peaufiné, millimétré et colporté à l'envi médias et réseaux sociaux. Le Gouvernement ne revient pas sur les mesures fiscales en faveur des plus riches, engagées en 2018 loin d'un tournant social, il s'agit davantage d'une pause tactique de votre part. Votre maître mot, dans la présentation de ce projet de budget, c'est la baisse des impôts. Présentée ainsi, l'affaire paraît séduisante. Cela signifie qu'il y aura mécaniquement moins d'argent dans les caisses de l'État, mais derrière une communication tonitruante se dissimule une tout autre réalité

Des milliards d'euros vont être accordés sans condition, alors que certains grands groupes continuent de délocaliser leurs usines à l'étranger, dans des pays à bas coûts de production. Ce nouveau cadeau pour le capital représente en fait 2,5 milliards d'euros en moins pour notre budget, nos hôpitaux, nos retraités, nos communes et le financement de la transition écologique. Ce n'est pas l'impôt qui est le problème, c'est l'injustice fiscale ; il faut la combattre. L'impôt donne à l'État les moyens de construire une société solidaire et juste. Je reprendrai à mon compte cette phrase d'Henry Morgenthau, secrétaire d'État au trésor du président Roosevelt dans les années 1930 : « Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Le consentement à l'impôt s'appuie sur des principes de justice fiscale, de progressivité et, surtout, sur l'idée que personne ne doit échapper à l'impôt, notamment les contribuables les plus importants. À ce propos, messieurs les ministres, nous sommes demandeurs d'informations détaillées sur la mission qui fut confiée à la Cour des comptes le 25 avril dernier par le Président de la République lors de sa conférence de presse clôturant le grand débat. Cette mission consistait en une évaluation du montant de la fraude et de l'évasion fiscales pour notre pays. Un rapport devait être rendu avant le débat budgétaire au Parlement. Le 2 décembre ! Nous sommes le 21 novembre, le texte arrive au Sénat et nous n'avons plus aucune nouvelle.

Oui, messieurs les ministres, ce sont bien les plus modestes qui subiront les effets de vos choix économiques et fiscaux. Votre baisse de l'impôt sur le revenu ne profitera évidemment pas à ceux qui ne gagnent pas assez d'argent pour être imposables. Vous proposez de faire des économies sur la santé, le logement, l'assurance chômage, les APL de nouveau, la vie étudiante et nos services publics de proximité. Vous avez fait le choix très libéral de vendre nos bijoux de famille avec la privatisation des groupes Aéroports de Paris et Française des jeux. Selon votre conception, pour que le travail paie, il faut passer par la caisse d'allocations familiales, avec la prime d'activité, par l'État, avec les baisses d'impôts, ou par la sécurité sociale, avec les allégements de cotisations. Bref, c'est à la solidarité nationale, c'est-à-dire à nous toutes et tous, de payer ces augmentations de salaires. On n'augmente pas vraiment les salariés, alors même que la distribution des dividendes bat encore des records cette année dans notre pays. Dans votre stratégie de communication, vous mettez en avant la restitution de pouvoir d'achat aux Français par le biais de la suppression de la taxe d'habitation. Cela est séduisant, mais il convient ici de bien analyser les conséquences de cette décision Cela vaut pour les communes, mais aussi pour les départements, qui ont clairement exprimé leur désaccord avec votre proposition de remplacer la taxe d'habitation des communes par la taxe sur le foncier bâti, perçue jusque-là par les collectivités départementales, d'autant que l'année de référence serait 2017 et non 2019. Lors du récent congrès de l'Assemblée des départements de France (ADF), les présidents de département, dans leur diversité politique, ont exprimé clairement leur opposition à cette mesure. De très nombreux départements connaissent déjà une situation financière très tendue. Ils considèrent aussi que les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les départements ne conservent pas de la liberté. C'est bien là une deuxième pierre d'achoppement, celle de l'autonomie financière des collectivités. Le projet de compenser les pertes par une part de TVA contrevient à ce principe : seul l'État a la maîtrise des taux de cette taxe, sans parler des aléas que le produit de celle-ci peut subir en fonction de l'intensité de la consommation, et donc de la croissance économique. Certes, on nous promet la compensation à l'euro près, mais les élus sont échaudés. Nous avons déjà entendu

comme l'urgence sociale, l'urgence climatique. Certes, on évoque une augmentation de 800 millions d'euros des crédits pour la transition écologique. Si Bercy a distribué un petit livret vert pour vendre ses actions, les choses ne bougent guère sur le fond.

Les besoins sont clairement identifiés. Il faudrait rénover 7 millions de logements qui sont de véritables passoires thermiques, au rythme d'au moins 700 000 logements par an. Nous en sommes aujourd'hui péniblement à 250 000, dont seulement 40 000 rénovations complètes. À l'évidence, nous prenons du retard. Sur la thématique des transports, il y a trop peu dans votre projet de budget pour investir massivement en faveur des transports ferroviaires, quasiment rien pour le fret, pour améliorer le transport des voyageurs avec davantage de dessertes et des billets moins chers. Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement serait bien inspiré d'accompagner les collectivités qui sont de plus en plus nombreuses à s'engager en faveur de la gratuité des transports collectifs. Le temps est venu d'une autre politique budgétaire, d'une autre logique de gestion. La réduction dogmatique de la dépense publique nous a conduits dans l'impasse. Il faut, messieurs les ministres, changer le logiciel de votre politique. Pour sortir de cette impasse, il aurait fallu s'attaquer aux près de 500 niches fiscales, qui représentent un total de 100 milliards d'euros. Le seul CICE, aujourd'hui transformé en baisse des charges patronales, aura coûté 100 milliards d'euros depuis sa création pour créer péniblement 130 000 emplois, nous dit-on. Vous n'annoncez rien de neuf en matière de lutte contre toutes les pratiques d'évitement de l'impôt toujours à l'oeuvre dans notre pays. Des dizaines de milliards d'euros échappent à la collectivité. C'est une lutte sans merci qu'il faut livrer contre ces pratiques scandaleuses. Il y a là des ressources abondantes à récupérer pour relever les grands défis de notre temps.

mais toutes les estimations disponibles montrent qu'en France les montants de la fraude sont très élevés. La multiplication des affaires prouve d'ailleurs que celle-ci se sophistique et qu'elle demeure extrêmement coûteuse. Il faut aussi relever que les effectifs du contrôle fiscal baissent depuis plusieurs années, ce qui se traduit par une baisse du nombre des contrôles et, par conséquent, par une baisse des résultats du contrôle fiscal : toujours cet écart saisissant entre une communication brillante et abondante et la réalité des choix faits par votre gouvernement de budget est très loin de répondre aux aspirations légitimes exprimées dans notre pays de manière de plus en plus marquée. Un budget, c'est l'outil de la justice sociale, de la justice fiscale et du progrès pour la société. M. Macron « président des riches », voilà une étiquette dont vous aurez du mal à vous débarrasser, à l'instar du fameux sparadrap du capitaine Haddock dans La parole est

Point de banqueroute. Point d'augmentation d'impositions. Point d'emprunts. Pour remplir ces trois points, il n'y a qu'un moyen. C'est de réduire la dépense au-dessous de la recette. Sans cela, le premier coup de canon forcerait l'État à la faillite. ces mots sont peut-être d'un autre siècle, mais ils ont gardé toute leur force. Ce sont ceux de l'illustre Turgot, dont Voltaire baisait les mains en pleurant. Ce sont les mots qu'il choisit pour présenter à Louis XVI son plan d'action destiné à restaurer la crédibilité de l'État face à la colère qui montait. Turgot n'eut que deux ans pour tenter d'assainir les finances ; Louis XVI crut bon de le congédier et céda de nouveau aux sirènes de l'emprunt et de la dette. Nous connaissons tous la suite. Nous ne sommes pas là pour parler d'histoire, mais une chose est sûre : quand les temps sont durs, et ils le sont aujourd'hui, deux années ne suffisent pas plus à vous, messieurs les ministres, qu'à Turgot pour assainir les finances publiques, et sans doute en France plus encore qu'ailleurs. encore qu'ailleurs. Nous devrons redoubler d'efforts, en 2020 et pendant de nombreuses années encore, pour pouvoir tirer définitivement un trait sur des années, voire des décennies, d'incurie budgétaire. Alors que nous commençons ce jour l'examen du projet de loi de finances pour 2020, il me semble judicieux de ne céder ni au triomphalisme ni au défaitisme. Car, à la vérité, si la situation s'améliore, c'est avant tout, comme dirait M. de La Palice, parce qu'elle a cessé de se détériorer. La barre des 100 % du PIB reste au-dessus de notre dette comme un bonnet d'âne au-dessus de nos têtes. Il faut d'abord reconnaître que le Gouvernement a repris le contrôle de la situation, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de dix ans. Les principaux voyants sont repassés au vert : la croissance économique poursuit son rythme tranquille, à 1,2 % du PIB, et elle se montre même résiliente aux tensions qui affectent le commerce international, tandis que la machine allemande, que l'on n'imaginait plus ralentir, commence à se gripper les prélèvements obligatoires sont contenus sous la barre des 45 % du PIB et le ratio de la dépense publique reflue légèrement à 53 % du PIB ; le déficit public s'établit à 2,2 % du PIB, nettement au-dessous de la barre des 3 %, dans les « clous » du traité Nous laissons derrière nous, comme un mauvais souvenir, la procédure européenne de déficit budgétaire excessif, dans laquelle notre pays s'était empêtré pendant des années. Nous étions nombreux sur ces travées à considérer que la maîtrise de notre déficit public constituait un préalable indispensable pour redorer l'image de la France sur la scène européenne et rassurer nos voisins quant à la fiabilité de notre modèle économique et social. C'est désormais chose faite, et le crédit en revient essentiellement au Gouvernement. Mais permettez-moi de ne pas m'en tenir à de bonnes paroles caoutchouteuses. En termes de déficit public, la France fait encore figure de mauvaise élève de la zone euro. Avec l'Espagne, l'Italie et la Belgique, notre pays a été épinglé par la Commission européenne, qui nous invite, dans son langage feutré, à « poursuivre des politiques budgétaires prudentes », et nous dit que la France présente- savourons la litote ! -« un risque de dérapage significatif de ses comptes publics par rapport aux ajustements requis ». nous rappelle enfin que bon nombre de nos partenaires ont su profiter d'un contexte macroéconomique favorable pour procéder aux ajustements nécessaires. Ce n'est pas encore tout à fait le cas de la France. Plus précisément, ce n'est pas le cas de l'État. Car le déficit public, cela a déjà été rappelé, est aujourd'hui exclusivement porté par l'État. Alors que les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale affichent des soldes excédentaires, et ce malgré l'imbroglio créé par le système des 35 heures, dont la débâcle des hôpitaux est emblématique, l'État reste dans le rouge. Le jour où les taux remonteront, nous risquons de redécouvrir ce que chacun sait bien dans sa vie quotidienne : les créanciers ont toujours une meilleure mémoire que les débiteurs. de budget de mi-mandat arrive enfin au Sénat. À la chambre des territoires, tous les regards sont rivés sur les réformes de la fiscalité locale. Nombreux sur ses travées sont ceux qui lisent entre ces lignes comptables comme un message d'alerte, et la bataille des chiffres n'a pas encore débuté que les communes craignent d'avoir déjà perdu la partie. Le groupe Les Indépendants veillera à ce que le grand jeu comptable ne se fasse pas aux dépens des communes, particulièrement pour ce qui concerne l'élaboration du déjà fameux « coco », le coefficient correcteur pour la compensation du transfert de la taxe d'habitation au budget de l'État.

comme le faisait remarquer le Président de la République avant-hier au Congrès des maires. Mais cela ne veut pas dire qu'ils comprennent, et qu'ils approuvent, le système qui la remplacera. Une chose est sûre : les Français font confiance aux maires, bien plus qu'au Gouvernement ou au Parlement, et ils ne veulent pas que les collectivités locales perdent au change. Nous y serons attentifs. Les collectivités locales, et singulièrement les communes, ont déjà fait leur part et dégagent maintenant des excédents budgétaires. Elles écoutent désormais l'État leur dire que tout va changer et qu'après tout ira mieux. Mais elles souhaiteraient qu'il réduise d'abord sa dépense publique, ou plutôt qu'il le fasse en même temps qu'il change la fiscalité locale. Certaines d'entre elles s'inquiètent de perdre la main sur une part importante de leurs recettes et de vivre un peu plus dans la dépendance de l'État. Dans cette optique, la question des valeurs locatives est loin d'être un détail technique. Si elles craignent de perdre sur le plan comptable, elles redoutent également de perdre sur le plan de l'autonomie fiscale. Je n'ignore pas les raisons qui conduisent le Gouvernement à de tels arbitrages. Vous avez mis le pouvoir d'achat au centre de votre politique économique, et vous avez le courage de conduire cette politique en réduisant la pression fiscale sur les ménages, notamment les plus modestes, sans laisser filer la dette, heureusement aidés par une conjoncture qui pourrait être plus mauvaise et des taux qui ne pourraient pas être plus bas. Dans cette optique, la baisse de l'impôt est une mesure salutaire. Le groupe Les Indépendants avait déjà proposé, l'an dernier, de baisser les taux marginaux sur les deux premières tranches du barème. Je me réjouis que vous ayez fait vôtre cette idée et je ne doute pas que le Sénat lui réservera cette fois un accueil favorable, car si la fable dit que le travail est pour les hommes un trésor, les Français commençaient à croire que l'État se l'accaparait ... Encore une fois, c'est la justice fiscale qui sous-tend les débats. Vous avez compris qu'il est indispensable, pour des questions de paix sociale, qu'en France le travail soit mieux rémunéré. Vous avez aussi compris que, pour la même raison, il est également indispensable que les impôts soient bien payés en France. C'est pourquoi notre groupe ne s'opposera pas à la domiciliation fiscale en France des dirigeants d'entreprises françaises, même si c'est les obliger plus que les inciter. Si je doute que cette mesure change la face du monde, elle aura le mérite, si précieux à notre époque, de faire comprendre que le fardeau du financement est équitablement partagé Je crois qu'il est ainsi possible de relocaliser et l'impôt et le travail. Tout ce qui simplifie la vie des entreprises sur le territoire national y contribue efficacement. C'est pourquoi nous soutiendrons également les mesures qui visent à supprimer progressivement les taxes à faible rendement et les niches fiscales, usines à gaz dont le coût de fonctionnement est en général inversement proportionnel à l'efficacité. Turgot, dans la même lettre adressée à Louis XVI, avait déjà identifié les obstacles que vous ne manquerez pas de rencontrer : « On demande sur quoi retrancher, et chaque ordonnateur, dans sa partie, soutiendra que toutes les dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons ; mais comme il n'y en a pas pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité absolue de l'économie. C'est inévitable : bien sûr, le Gouvernement sera systématiquement critiqué lorsqu'il supprimera en même temps des recettes et des dépenses. Quoi qu'il fasse, on préférerait toujours qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. L'année qui s'est écoulée en a apporté une nouvelle fois la preuve. Les formes changent, mais le fond demeure le même : les Français aiment l'État qui donne et détestent l'État qui prend, et ils refusent souvent de voir que ce sont les deux faces d'une même médaille. Comme dans beaucoup de pays, l'État est vécu, non parfois sans quelque raison, comme un monstre à deux bras inégaux, un très long bras pour prendre et un bras très court pour donner. Mais ces critiques ne doivent pas ôter le courage d'aller de l'avant en matière d'équilibre budgétaire. Oscar Wilde disait que le mariage est la principale cause de divorce. On peut dire de la même façon que la dépense publique est la principale cause des impôts, et tout le reste est un mensonge sur lequel finit toujours par germer la haine d'un autre fantasmé, des responsables politiques aux riches, en passant par les chômeurs et les étrangers. Alors que, à la veille du 5 décembre, il est plus difficile de trouver en France un esprit tranquille qu'un trèfle à quatre feuilles, le Gouvernement doit composer avec une urgence plus grande encore que la réduction de la dette publique non contents de devoir déjà réduire drastiquement notre dette publique, nous devons maintenant, et de toute urgence, réduire notre dette climatique. Vous avez pris le sujet à bras-le-corps, sans céder à la démagogie qui consiste à faire croire que les finances ne comptent pas face au climat. la température sont devenus le nouveau prétexte de ceux qui veulent apporter à ce problème aussi immense qu'inédit la vieille solution de la dépense publique. On entend dire, çà et là, qu'il faudrait exclure de l'application des critères de Maastricht toutes les dépenses qui contribuent à la transition écologique. On comprend bien l'intention, et l'on serait tenté d'accepter si la méthode ne ravivait pas quelques mauvais souvenirs : il faudrait alors mettre en place un comité central de planification écologique qui déciderait, depuis le 139 rue de Bercy, ce qui rentre ou non dans les clous de la révolution écologique, comme le prône le de la France soumise à Cuba ! La vérité, c'est que l'urgence climatique nous met face à nos contradictions. Chacun sait qu'il nous faudra renoncer à notre confort et redoubler d'efforts pour être à la hauteur des enjeux. Mais je pense que nous saurons trouver là le moyen de nous élever collectivement. Nous savons tous qu'il n'y a aucune alternative. Dette climatique, dette publique, même combat. Et dans les deux cas, il faut de la rigueur. Rappelons-nous le mot de Paul Valéry : « La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. Les mesures de fiscalité écologique que vous proposez vont dans le bon sens. Elles se focalisent sur les deux secteurs qui contribuent le plus aux émissions de CO2 en France, à savoir le logement et le transport, part, du soutien aux travaux de rénovation énergétique, et, d'autre part, de la diminution des avantages fiscaux pour les carburants fossiles. Cette approche réintroduit un peu de rationalité dans les débats et est plus progressive. Nous la soutiendrons. Il est toujours plus confortable d'imaginer que la seule solution pour s'adapter aux temps modernes consiste à faire table rase du passé, mais c'est souvent la pire erreur que d'oublier le monde d'hier pour penser le monde de demain. C'est pourquoi la réduction de notre dette publique doit être menée parallèlement à notre transition écologique. Il faut solder les comptes sans chercher à tout prix à désigner des coupables. D'aucuns disent que les réformes ne vont pas assez vite pour réduire en même temps notre dette publique et notre dette climatique. Je crois qu'elles vont tout de même dans la bonne direction. La parole

quand bien même il fallait, pour cela, s'écarter des objectifs initiaux de la loi de programmation des finances publiques. En effet, derrière l'impôt auquel nous consentons, derrière la dépense que nous autorisons, c'est l'humain qui doit guider notre action, et non pas seulement les ratios financiers. Bien sûr, nous devons conserver l'objectif du redressement des comptes publics ; nous y tenons, car c'est ainsi que nous préparons l'avenir ; mon collègue Vincent Delahaye reviendra sur ce sujet. Mais ne nous trompons pas sur les moyens d'y parvenir : nous ne réussirons pas le redressement des finances publiques s'il ne s'accompagne pas d'une politique efficace de réduction des inégalités. Comment pourrait-on aujourd'hui continuer à courir derrière une baisse drastique et toute théorique du nombre d'agents publics alors que nous avons besoin de plus de personnel hospitalier, que nous devrons relever le défi de la dépendance, que nous avons besoin d'enseignants et d'accompagnants dans nos écoles, de davantage de policiers et de gendarmes pour mieux répondre à la menace terroriste ? Et on pourrait continuer la liste ! Même si, évidemment, des des réorganisations et des redéploiements sont nécessaires, même si des réductions d'effectifs et des économies sont possibles, notamment dans les agences et autres organismes satellites de l'État,

depuis le début de l'année, 5,6 milliards d'euros ont été recouvrés par l'État au titre de la lutte contre la fraude fiscale, soit 40 % de recettes en plus par rapport à l'an dernier. Sur ce terrain, de nombreuses pistes encore à explorer : vous en avez évoqué quelques-unes, et ma collègue Nathalie Goulet reviendra sur ce sujet, sur lequel elle a beaucoup travaillé. Ce projet de loi de finances doit finalement tenter de respecter un difficile équilibre, en tenant compte de la réalité sociale et en répondant aux enjeux auxquels est confrontée notre société sans pour autant perdre de vue le nécessaire redressement des comptes publics. Le déficit public, établi à 2,2 % du PIB, est certes encore élevé, mais il est à son niveau le plus faible depuis vingt ans, et ce malgré une baisse historique des prélèvements obligatoires, à hauteur de 9 milliards d'euros. Voilà la réalité La justice fiscale sort renforcée de la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu au profit des premières tranches d'imposition. Nous saluons également la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le taux devrait Enfin, l'article 5 entérine la suppression de la taxe d'habitation en 2020 pour 80 % des ménages et en 2023 pour les 20 % restants. Quel que soit l'avis que l'on porte sur le bien-fondé de cette mesure, la réalité est qu'elle induira un gain de pouvoir d'achat moyen de plus de 700 euros par ménage concerné. Ce projet de budget donne également le coup d'envoi de la réforme de la fiscalité locale, suivant des modalités finalement assez proches de celles qu'avait proposées la commission des finances du Sénat en 2018. La question du mode de compensation a suscité beaucoup d'inquiétude chez les élus, une inquiétude justifiée au regard des plus de 2 milliards d'euros perdus chaque année par le seul bloc communal du fait des mécanismes de compensation inadaptés institués lors des précédentes réformes. C'est pourquoi nous approuvons le principe général proposé, qui vise à substituer au produit de la taxe d'habitation perdu, pour chaque niveau de collectivité, une nouvelle recette fiscale, ce qui leur garantira une ressource pérenne et dynamique.

que l'attribution d'une part de l'impôt national qu'est la TVA a un effet péréquateur qui préservera les départements les plus fragiles. Je sais que les avis divergent sur cette question, mais, élu du Cantal, je connais parfaitement les limites de l'autonomie fiscale, tant recherchée

de 180 millions d'euros pour les communes, et la réforme de la péréquation entre départements, d'ailleurs voulue par les départements eux-mêmes, renforcent la solidarité en faveur des collectivités les plus fragiles. est présenté devra néanmoins être corrigé sur plusieurs points d'importance. D'abord- c'est le point essentiel à mes yeux -, le risque d'une variation du potentiel financier de l'ensemble des collectivités sous l'effet de la réforme de la taxe d'habitation devra impérativement être écarté. C'est un risque majeur de cette réforme à forte incidence sur le niveau des dotations. Sans mécanisme de neutralisation,

un mécanisme de garantie dans le temps des recettes des départements devra être mis en place pour sécuriser leurs ressources sur la durée. Il faut conclure, mon cher collègue. Quelques points saillants restent donc en suspens : notre groupe contribuera activement au débat

Merci

Le « ni oui ni non » britannique sans fin sur le Brexit, les postures de puissance de certains dirigeants qui alimentent des conflits commerciaux, l'impact des crises au Moyen-Orient sur les cours des hydrocarbures, tout cela pèse défavorablement sur la croissance mondiale. croissance mondiale. MM. les ministres l'ont rappelé, ces tensions coûteront probablement 0,5 point de croissance en 2020. Malgré ces conditions difficiles, gardons le cap pour imprimer à notre politique budgétaire, autant que

Aussi la réduction du déficit public doit-elle être poursuivie. Le retour sous la barre des 3 % du PIB est heureusement intervenu dès 2017, et la perspective d'un déficit ramené à 2,2 % du PIB est réjouissante, même si elle est en deçà de la cible prévue par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Quant à la dette publique, elle décroît très légèrement : c'est bien, mais ce n'est sans aucun doute pas assez, malgré le renfort de taux d'intérêt très bas. On connaît les conditions de ces dérapages pour l'exercice budgétaire 2019 : ils sont en partie la conséquence des mesures adoptées en réponse à la crise des « gilets jaunes C'est la difficulté de tout exercice budgétaire : pouvoir digérer les aléas, qu'ils soient sociaux ou économiques. Il est donc important de retrouver des marges en faisant fondre au plus vite notre déficit structurel. En attendant, afin d'éviter l'éventuel retour de colères contenues, qui coûterait encore très cher, tentons de mettre en oeuvre la politique la plus équitable possible. Des mesures de soutien en direction des ménages les plus modestes ont été adoptées l'année dernière ; le RDSE les avait très largement approuvées. Cette année, le projet de budget cible également les classes moyennes, avec une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros qui les concernerait. C'est une bonne chose, mais l'équité passe aussi par un certain ménage fiscal.

L'équité est aussi un principe qui doit prévaloir à l'égard de nos entreprises. Est-il normal que le commerce physique ait été imposé à hauteur de 47,3 milliards d'euros en 2018, tandis que la contribution fiscale des GAFA s'établit à seulement 67 millions d'euros ? Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes très sensible à cette problématique. Trois articles du présent projet de loi de finances ciblent particulièrement l'e-commerce. Pour aller plus loin, je proposerai d'assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les entrepôts des plateformes en ligne, les. Rappelons Rappelons que le commerce physique représente 2,8 millions d'emplois ; à ce titre, il contribue très largement à la croissance de notre pays et au dynamisme de ses territoires. J'en viens au troisième principe qui doit sous-tendre le budget de l'État : l'efficacité, au service de nos entreprises, mais aussi de nos collectivités locales. Je salue le maintien de l'objectif de baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le taux devrait

du crédit d'impôt recherche. À reprendre d'une main ce que l'on donne de l'autre, on risque de gripper la politique de l'offre alors que clignotent des signaux de ralentissement économique. Aussi proposerai-je quelques amendements portant sur deux secteurs importants pour notre économie : les opérateurs de télécommunications et l'aviation civile. Pour le premier, une certaine modération fiscale serait souhaitable,

exponentiel. Concernant le secteur du transport aérien, le pavillon français s'emploie à relever les défis environnementaux, dont celui de réduire de 50 % ses émissions de CO2 à l'horizon 2050. Dans un contexte de forte concurrence internationale, je proposerai quelques mesures visant à soutenir les compagnies dans leur transition écologique et à alléger le poids fiscal du dispositif de l'article 20, qui pèse sur elle.

en ce qu'elles apportent des réponses de proximité très opportunes, grâce leurs capacités d'investissement. Néanmoins, malgré toute la bonne volonté des élus, leur efficacité dépend là aussi

quand elles voient une régression de leurs ressources à hauteur de 120 millions d'euros. Vous voyez une neutralité de la suppression de la taxe d'habitation, quand elles craignent un impact à court terme. Qu'en est-il en réalité ? Le Sénat, soucieux des collectivités locales qu'il représente, attend des garanties

D'où vient le sentiment, assez général en France, d'une forme de paupérisation, au-delà de cette statistique ?

alors que le débat politique de ces dernières semaines a parfois été occulté par des sujets de société qui, s'ils ont indubitablement leur importance, ne concernent parfois que très indirectement nos concitoyens, il est temps d'engager la discussion au fond de ce projet de loi de finances pour 2020. Davantage que les polémiques suscitées par des entretiens accordés à, ce sont les débats que nous entamons qui permettront de jauger l'action concrète du Gouvernement pour nos concitoyens, dans un contexte où les attentes sont grandes et- permettez-moi de le dire, monsieur le ministre -légitimes eu égard aux résultats décevants, pour ne pas dire plus, du Gouvernement à ce jour. Mes chers collègues, ce qui prime, ce sont les dépenses engagées par le Gouvernement depuis le début de cette mandature. Néanmoins, au groupe socialiste et républicain, nous demeurons convaincus

Votre gouvernement a d'ailleurs, monsieur le ministre, placé la barre très haut en la matière en début de quinquennat, avec beaucoup d'aplomb. Claude Raynal et moi-même avons retracé vos prévisions budgétaires, entre la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,

C'est aujourd'hui sur un déficit de 1,5 % que vous tablez. Vous nous promettiez, à l'époque, une dette publique s'élevant à 91,4 % du PIB. C'est aujourd'hui sur une dette atteignant 97,7 % du PIB que vous tablez. Vous nous promettiez également alors une dépense publique limitée à 50,9 % du PIB. C'est aujourd'hui sur une dépense de 52,3 % du PIB que vous tablez. Permettez-nous, monsieur le ministre, de douter de la crédibilité de vos annonces récentes devant notre commission des finances.

Certes, vous invoquerez la récession internationale, la crise des « gilets jaunes », vous vous targuerez de meilleurs résultats que nos voisins européens, voire que vos prédécesseurs.

la croissance moyenne était de 0,36 % et le déficit a progressé de 1,4 %, alors que la France traversait la crise économique la plus dure de ces trente dernières années. Chers collègues de la majorité sénatoriale, nous reconnaissons que la conjoncture économique était peu porteuse à l'époque ! Il est temps ! Durant le quinquennat Hollande, la croissance moyenne était de 1,07 % et le déficit a chuté de 2 points. Pour le moment, avec une croissance largement supérieure, de 1,68 % en moyenne, vous avez réussi l'exploit de réduire le déficit de 0,6 % ! Je ne crois pas que cela puisse légitimer les leçons que le Gouvernement se plaît à adresser à l'« ancien monde l'équilibre budgétaire n'est pas, il est vrai, la fin en soi d'une politique budgétaire. Au vu de ces renoncements, nous aurions pu nous attendre à ce que nos concitoyens bénéficient d'un réel effort de la part d'un gouvernement qui s'est illustré jusqu'à présent par son souci de protéger les grands groupes et les plus aisés. Nous avons cherché, dans ce projet de loi de finances pour 2020, mais nous n'avons rien trouvé. Certes, il y a eu les mesures « gilets jaunes », qui, soit dit au passage, ont coûté à l'État deux fois plus que le montant des économies qu'il comptait réaliser au travers du projet de loi de finances pour 2020. Certes, il y a les 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu, monsieur le ministre, pour être exhaustif, pourriez-vous nous rappeler à combien se chiffre la hausse des recettes fiscales et non fiscales de l'État consécutive notamment à l'adoption du prélèvement à la source, que nous avons engagée sous le précédent gouvernement et soutenue sous le vôtre ? avait été proposée par le précédent gouvernement. Même quand vous tentez, sous la contrainte, de mettre en oeuvre une politique à destination de certains de nos concitoyens qui en ont besoin, vous déployez des trésors d'inventivité pour en annuler la portée. Je me permets de rappeler que près de 5 millions de foyers n'ont pas vu la couleur de la suppression de la taxe d'habitation

Que proposez-vous de concret pour mettre en oeuvre la transition écologique ? Malgré des recettes supplémentaires et la modestie de la redistribution, vous n'arrivez même pas à équilibrer vos comptes

somme, vous reprenez d'une main ce que vous avez donné de l'autre. Monsieur le ministre, je me permets une suggestion : le rétablissement de l'ISF, que nous vous avions proposé et que nous vous proposerons de nouveau, aurait permis de dégager des recettes fort opportunément pour répondre aux besoins et à la demande de plus de justice fiscale. Oui ! C'est sûr ! En effet, le rapport du président Vincent Éblé et du rapporteur général Albéric de Montgolfier a permis d'établir que le gain moyen lié à la mise en place de l'IFI a été, pour les 100 premiers redevables de l'ISF au titre de 2017, de 1,2 million d'euros par foyer. Nos propositions de bon sens, de justice fiscale et les alertes du Sénat auraient dû vous faire entendre raison. Qu'attendez-vous ? Que les mouvements sociaux du 5 décembre dégénèrent ? Cette posture de pompier pyromane qui est la vôtre ne vous honore pas et elle est dangereuse. Pour conclure, le groupe socialiste et républicain souhaite tendre la main au Gouvernement et à la majorité sénatoriale. Nous avons publié, voilà quelques semaines, un contre-budget qui témoigne, si besoin était, de la crédibilité d'une autre orientation politique que celle que vous avez choisie.

de juillet dernier, à l'occasion de la signature des premiers contrats de convergence et de transformation entre l'État et les outre-mer, le Président de la République a rappelé le principe de base guidant sa politique pour nos territoires ultramarins en déclarant haut et fort que l'« on ne fait pas d'économies sur les outre-mer ». ». Je dois dire que le Gouvernement a respecté la parole présidentielle. L'examen du projet de budget de la mission « Outre-mer » fait apparaître une stabilité des crédits de paiement, à 2,358 milliards d'euros, la baisse apparente étant due, pour l'essentiel, à des mesures de périmètre, pour 100 millions d'euros, et, pour 34 millions d'euros, à la compensation moindre des exonérations de charges sociales. On s'en rend encore mieux compte en considérant, toutes missions confondues, l'ensemble des crédits consacrés aux outre-mer, la mission « Outre-mer » ne représentant finalement que 11,6 % du total.

dans l'« archipel France », il y a des îlots de pauvreté et de précarité, des îlots en retard de développement, que nous n'arrivons pas à résorber. Ainsi, le PIB par habitant de la Guyane est de 14 800 euros, inférieur de moitié à celui de la métropole. Pis, celui de Mayotte est à peine de 9 100 euros. Malgré les moyens engagés, les situations sont telles en outre-mer que cela semble toujours insuffisant.

D'après les données pour 2018 d'Eurostat, 21,3 % des jeunes Ultramarins âgés de 18 à 25 ans quittent prématurément le système d'éducation et de formation. En corollaire, le chômage des jeunes, qui s'établit à plus de 40 %, continue d'augmenter. Le défi que lance cette jeunesse est énorme. Pour le relever, les crédits consacrés à l'éducation et à la jeunesse augmentent de plus de 200 millions d'euros en deux ans, sans compter le maintien de dotations spéciales, pour un montant de 90 millions d'euros, à destination des collectivités de Guyane et de Mayotte afin d'aider à la construction d'établissements scolaires. Divers dispositifs sont par ailleurs renforcés au travers de ce PLF, comme le service militaire adapté, dont les capacités d'accueil sont portées à plus de 6 000 jeunes. de juillet 2019, la signature de contrats de convergence et de transformation entre les collectivités régionales et l'État, pour un montant de 2,1 milliards d'euros sur quatre ans, est venue concrétiser la volonté du Gouvernement de mener une politique véritablement à la hauteur des enjeux ultramarins. Leur traduction dans ce PLF confirme cet engagement. Cependant, ce que je souhaite souligner avec force aujourd'hui, c'est que ce projet de loi de finances pour 2020 reconnaît pour la première fois l'iniquité de traitement entre les collectivités locales d'outre-mer et celles de métropole. Cela fait des années que les collectivités ultramarines sont sous-dotées en matière de péréquation, et des années que j'en fais le constat sans être entendu. Il en est désormais autrement. Le Gouvernement a chiffré l'écart, pour les communes d'outre-mer, à 85 millions d'euros, qu'il propose de rattraper sur cinq ans. Permettez-moi tout de même d'exprimer ma déception de voir que la commission des finances a préféré s'aligner sur la position du Comité des finances locales en proposant un amendement visant à augmenter le montant total de la DGF, très certainement pour ne pas brusquer les communes de l'Hexagone. Cet amendement montre à quel point la solidarité n'est pas encore une valeur partagée par tous. Pour autant, il faudra plus qu'une augmentation de dotation pour sortir de l'ornière financière

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'équilibre, c'est la santé, y compris en matière budgétaire. Oui ! Ce n'est un scoop pour personne ici : la France fait partie des derniers pays de la classe européenne en matière de déficit.

Je veux parler de l'Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas, de la République tchèque. Pour moi, tout est lié : santé budgétaire, santé économique et santé sociale. santé sociale. Pour lutter contre le chômage et l'inactivité, faut-il toujours plus de dépense publique et plus de déficit ? Je pense l'inverse : il faut moins de dépense publique et moins de déficit.

! Comment revenir à une situation saine ? Faut-il augmenter les impôts ? Il y a déjà overdose ! Pour revenir à l'équilibre budgétaire, il faudrait, sur une seule année, augmenter tous les impôts, y compris la TVA et la CSG, de 33 %.

Les 35 heures de Martine Aubry ont fait beaucoup de mal à notre économie, et pas seulement à l'hôpital. Nous sommes le pays où l'on travaille le moins, avec un taux de chômage très élevé. Le partage du temps de travail a totalement échoué, mes chers collègues.

L'an passé, à la même période, les Français se mobilisaient sur les ronds-points, comme en écho à nos avertissements. Votre refus d'écouter la voix du Sénat et un certain entêtement auront fait perdre des mois d'action précieux à la France, au prix de vives tensions sociales, jamais vues sous la V République. Après de telles crispations, nous aurions pu croire la leçon retenue. Nous aurions pu croire que les appels à garantir la traçabilité de l'utilisation des recettes de fiscalité énergétique avaient été entendus.

l'an dernier. L'augmentation massive, brutale et aveugle de la trajectoire carbone a pris de court et à revers, dans un contexte de hausse du prix des carburants, des milliers de Français, souvent automobilistes, assignés à résidence et

C'est une grave erreur : ce sujet devrait, tout au contraire, rassembler nos concitoyens pour « faire France » ensemble. Il y a pis encore. Avec l'arrêt en rase campagne de la trajectoire carbone, vous ne disposez plus de la fiscalité énergétique pour financer vos plans de sauvetage. je vous reconnais un certain don d'inventivité : lorsqu'il n'est plus possible d'augmenter les recettes écologiques, vous baissez les dépenses traduit votre volonté de vernir une fiscalité de rendement en prétendant la verdir ... Vous êtes en fait de faux dévots de l'écologie, de vrais tartuffes verts.

tartuffes quand vous prétendez faire de l'éco-contribution sur les billets d'avion une mesure écologique : vous impactez en fait notre compagnie nationale et, surtout, la taxe financera la réparation des radars routiers détruits l'année dernière tartuffes, enfin, en matière d'utilisation des recettes issues de la fiscalité verte, quand vous supprimez les comptes d'affectation spéciale écologiques, qui permettent la traçabilité de l'emploi de ces recettes. Messieurs les ministres, ce projet de budget porte également la marque de vos renoncements renoncements : renoncement à proposer une nouvelle fiscalité environnementale, juste, adaptée et accompagnant les Français ; renoncement à investir dans la transition énergétique,

Alors, comme on sort un lapin du chapeau, vous dégainez ce livre vert, succédané peut-être du petit Livre rouge. Tout cela, mes chers collègues, ce n'est pas un acte II plus vert, une nouvelle étape, c'est du. Quant

Pourtant, le temps presse. D'une part, qu'il s'agisse du climat ou de l'équilibre de nos finances publiques, vous hypothéquez l'avenir de nos concitoyens. Présenter un budget financé massivement par la dette, lorsque celle-ci représente déjà près de 100 % de notre richesse nationale, c'est jouer avec le feu.

évoquent une convergence des luttes ou en rêvent exposent la France à une coalition des colères. Les semaines passent, et les revendications s'accumulent chez les agriculteurs, chez certaines de nos forces de sécurité et de protection, chez les enseignants, chez les personnels de santé et les personnels soignants, chez les étudiants ... Messieurs les ministres, je ne veux pas souffler sur les braises, mais je tiens à vous dire que le pays ne peut demeurer dans cet état de tension permanente. À trop laisser couver le feu sous la cendre, vous risquez l'incendie. Je crois bon de rappeler que la vraie chambre de refroidissement, le lieu de l'apaisement, c'est le Parlement. Personne ne gagnera à voir se multiplier les revendications dans la rue, suivies d'annonces médiatiques ou de plans de sauvetage, toujours financés par la dette. Face à de telles tensions, il est urgent de renouer avec les Français, par le biais de leurs représentants, un contrat démocratique qui soit un pacte écologique, social et économique. Le débat démocratique doit se tenir au Parlement. C'est dans nos assemblées que doivent se dire la vérité des chiffres, s'élaborer le diagnostic partagé et se dessiner la feuille de route commune pour la maison France.

comme celui de l'acte II du quinquennat, censé être marqué par une baisse massive d'impôts et s'inscrivant dans un contexte « de croissance française robuste Mais derrière la communication, la croissance est en réalité bien fragile, et largement due aux mesures d'urgence prises par le Gouvernement à la suite du mouvement des « gilets jaunes

Prenons même la suppression de la taxe d'habitation, qui était censée garantir une fiscalité plus juste pour les Français : en réalité, les 5 millions de foyers les plus modestes, qui ne la payaient pas, ne bénéficieront donc pas de sa suppression. ! À l'inverse, les 20 % de Français les plus favorisés feront un gain de 8 milliards d'euros, soit autant que les 80 % des Français appartenant à la classe moyenne. Ainsi, la suppression de la taxe d'habitation, présentée lors de la campagne présidentielle comme une mesure de justice sociale,

Par ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, la suppression de la taxe d'habitation ne sera pas intégralement compensée aux communes, puisque 250 millions d'euros leur manqueront, ainsi qu'aux intercommunalités, dès 2020.

les grands perdants des mesures fiscales du Gouvernement sont les 25 % de Français les plus modestes, particulièrement les 10 % de ménages les plus pauvres. Si l'on ajoute le fait que le fait que ces foyers les plus modestes ne bénéficieront ni de la suppression de la taxe d'habitation ni de la baisse de l'impôt sur le revenu, il apparaît clairement qu'ils sont de nouveau les grands perdants. En valeur absolue,

vous ne renoncez pas plus en 2020 qu'en 2019 ou en 2018, ce qui vous conduit d'ailleurs à conserver un déficit budgétaire important sans pour autant financer les actions publiques dont notre pays a besoin.

Quel signe de volontarisme ... Avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, nous ne pouvons pas nous retrouver dans un projet de budget qui ne permet ni la justice sociale, ni la transition énergétique,

ni même de réduire les déficits publics au rythme annoncé en débat de quinquennat ! Quelle caricature ! Manque de justice, manque d'ambition, manque d'efficacité ... Depuis un an, tout a changé, mais, en réalité, rien n'a changé. Voilà pourquoi, au-delà

pour examiner le projet de loi de finances pour 2020, il convient de le replacer dans un contexte international toujours aussi incertain et sans doute encore plus perturbé qu'il y a un an. La multiplication des conflits et des contestations dans le monde, l'attitude agressive des États-Unis dans ses relations commerciales avec la Chine, l'Europe, en particulier la France, feuilleton du Brexit et le manque de cohésion des pays européens ne sont pas de nature à nous rassurer et constituent une toile de fond peu propice aux investissements et aux initiatives. Ce tableau est encore assombri par nos propres insuffisances économiques, notamment la persistance d'un déficit du commerce extérieur supérieur à 50 milliards d'euros, avec un secteur industriel affaibli qui a du mal à retrouver sa place de moteur de la croissance. Au-delà du contexte, des hypothèses macroéconomiques et des grands équilibres financiers, ce projet de budget présente de nombreuses mesures fiscales qui, pour certaines, reprennent des engagements de début de mandat, et, pour d'autres, constituent des nouveautés. Par ailleurs, le Gouvernement poursuit, en seconde partie du PLF, la trajectoire de renforcement des grandes missions régaliennes- défense, justice, sécurités -ou d'éducation et d'investissement- enseignement, recherche, investissements d'avenir. En termes de grands équilibres, le déficit diminue pour s'établir à 2,2 % du PIB. En réalité, cela correspond à un niveau identique à celui de 2019 si l'on retire, pour cette année-là, le double effet de la transformation du CICE en allégement pérenne de cotisations sociales. Pour sa part, le niveau de la dette publique est également quasiment stable, à 98,7 % du PIB. Il n'y a donc pas d'amélioration structurelle des comptes publics, avec un déficit qui dépassera encore 90 milliards d'euros. cette apparente stabilité ne doit pas masquer les efforts accomplis pour faire face à une situation conjoncturelle compliquée, avec de multiples sollicitations sectorielles et une protestation sociale symbolisée par la crise des « gilets jaunes », que l'on invoque un peu trop fréquemment pour

a conduit le Gouvernement, avec, pour l'essentiel, l'accord du Parlement, à mettre en oeuvre un ensemble de mesures d'un coût budgétaire de l'ordre de 17 milliards d'euros, principalement pris en charge par le budget général et, partiellement, par celui de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il semblait évident que la trajectoire des finances publiques pour 2018-2022 subirait un léger infléchissement, reportant dans le temps le rétablissement complet de l'équilibre budgétaire. Le budget de 2019 et celui de 2020 ont ainsi montré leur capacité d'absorption de charges nouvelles non programmées, allant du renforcement de certaines prestations à des diminutions de recettes fiscales, en passant par des compensations de la suppression d'impôts locaux ou par la prise en compte de charges externes, externes, comme les intérêts d'emprunt liés à la reprise progressive de la dette de la SNCF. Bien entendu, cette politique « temporairement de la demande » a des effets positifs sur la TVA, par un sursaut de consommation,

le projet de budget pour 2020 nous inspire un certain nombre de satisfactions, mais aussi quelques interrogations et inquiétudes. Commençons par ces dernières. On constate un effort significatif de l'État en direction des entreprises, qui ne se traduit pas encore de de manière importante sur la croissance, l'emploi et le commerce extérieur, une insuffisance marquée des efforts pour réduire la dépense publique, en particulier dans le périmètre de l'État-

Parmi les satisfactions, on relève une grande sincérité des comptes, fondés sur des prévisions de croissance du PIB jugées crédibles et une certaine prudence des estimations. Je pense notamment

Je voudrais également évoquer les relations avec les collectivités locales. Les concours qui leur sont accordés sont stabilisés, avec une enveloppe de l'ordre de 40 milliards d'euros. Après des années de baisse des dotations, cette situation peut être considérée comme satisfaisante. Nous ne doutons pas non plus que la suppression de la taxe d'habitation sera compensée à l'euro près pour les communes. En revanche, cette dernière mesure a pour principal inconvénient de couper le lien financier entre une partie des habitants et la collectivité mettant en place les services qui leur sont destinés. Cette suppression, compensée par le fléchage d'une fraction de TVA, aura des conséquences sur tout le dispositif fiscal et de dotations de l'État en direction des collectivités, ce qui sera peut-être l'heureuse occasion d'une remise à plat complète.

C'est une stratégie qui, structurellement, peut fragiliser le budget de l'État. Il conviendrait peut-être de ne pas l'étendre, à l'avenir, à d'autres dispositifs de compensation. Sur le détail des mesures par mission, la majorité du groupe RDSE n'entend pas s'opposer aux orientations définies par le Gouvernement, mais elle souhaite que soient adoptées, par voie d'amendements,

encore, il me revient de parler du sort réservé aux collectivités territoriales dans le projet de loi de finances. La situation n'est pas meilleure qu'à l'automne 2018. À mon sens, l'État devrait largement s'inspirer de leur rigueur de gestion.

vous communiquez en parlant de baisses d'impôts, en alimentant une confusion entre les différents types de prélèvements- cotisations, impôts et taxes -et leurs effets, très différents sur le plan redistributif Cette confusion atteint son paroxysme cette année avec l'officialisation de la non-compensation des baisses ou des exonérations de cotisations sociales que vous décidez. On la retrouve dans l'exonération de taxe d'habitation, le transfert de la taxe foncière des départements aux communes et sa compensation l'attribution d'une part de TVA. L'argument le plus utilisé pour justifier ce choix consiste à mettre en avant le côté « dynamique » de cet impôt. Notre croissance reposant essentiellement sur la consommation des ménages, nous avons effectivement un impôt indirect dynamique, mais ô combien injuste ! Il faut le rappeler sans relâche, la TVA est l'impôt le plus injuste.

50 euros pour ces chaussures, 10 euros pour le Trésor public ; 10 000 euros pour cette voiture, 2 000 euros pour le Trésor public ! Je vous l'assure, nous parlerions beaucoup moins dans cet hémicycle de l'impôt sur le revenu que de la TVA, et les Français nous demanderaient de baisser cette dernière

pour financer des baisses de cotisations patronales. Aujourd'hui, c'est par la petite porte des baisses de cotisations que nous voyons introduire cette TVA sociale. Cela se fait à bas bruit, lentement mais sûrement, en fléchant vers la compensation partielle à la sécurité sociale une part plus importante de la TVA.

Le projet consistant à transférer la taxe foncière des départements vers les communes et les EPCI en compensant ce transfert par l'attribution d'une part de la TVA est l'étape suivante de la création d'une TVA territoriale. Cela accentuera les injustices territoriales.

que la TVA est aussi éminemment injuste. TVA sociale, TVA territoriale : la baisse de l'impôt sur le revenu cache une aggravation de l'injustice fiscale dans notre pays. En outre, la baisse de l'impôt sur le revenu, qui a été rendue possible par une meilleure perception de l'impôt à la source, est présentée comme une mesure en faveur du pouvoir d'achat. C'est vrai pour beaucoup de Français,

M. Macron, dans du 8 novembre dernier, découvrait que les investissements d'avenir ne devraient pas entrer dans le calcul du déficit et que la rigueur budgétaire, organisée autour de la règle des 3 % de déficit, était d'un autre siècle. Peut-être devrions-nous le prendre au mot, notamment quand il s'agit de financer les dépenses d'investissement essentielles en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Six ans plus tard, le temps ayant fait son effet, elle se trouve toujours sous surveillance, mais, cette fois, pour dette excessive. Et le commissaire européen de le rappeler : « L'absence d'effort structurel implique la stabilisation de la dette à des niveaux très élevés. » La remarque est cocasse quand on songe à son action, cruelle quand on songe à la vôtre

dans le fracas des marches forcées des « gilets jaunes ». Vous avez préféré baisser des impôts qui ne sont pas les vôtres, comme l'a rappelé de manière cinglante François Baroin : ceux des collectivités ou encore ceux qui créent la dette que paieront nos enfants, comme l'a souligné Bruno Retailleau. Pourtant, et il faut s'en réjouir, la conjoncture économique vous aidait, avec des taux d'intérêt négatifs, des rentrées fiscales liées à votre réforme bien menée - il faut le reconnaître, monsieur le ministre -du prélèvement à la source ... Le Sénat était contre Cette embellie conjoncturelle est votre alibi pour l'absence d'efforts structurels : aucune réduction du déficit structurel en 2020, comme le souligne le très neutre Haut Conseil des finances publiques.

ni l'État ni la sécurité sociale que vous régissez par la loi ne sont au rendez-vous de cette programmation pluriannuelle. Pas de cap, et plus de limites,

Pas de cap tout court : votre capitaine a perdu la boussole, vous naviguez à vue alors que le bateau des administrations publiques prend l'eau de toutes parts. Vous croyez colmater les fuites en déplaçant l'eau dans la cale vite, récupérons la dette de la SNCF ! Vite, récupérons celle des hôpitaux, mais laissons aux départements la dette sociale que l'État a omis de compenser ! C'est un bateau ivre, livré à des réalités bien moins poétiques. Votre politique des finances publiques est illisible, et donc inacceptable, car quel peut être le consentement à l'impôt lorsque tout part en tuyauterie ?

Plus de cap ni de bon sens ! À la sécurité sociale, des cotisations qui ouvrent des droits ; aux collectivités, des impôts à base locale pour que les élus rendent réellement des comptes, car, comme le rappelle Gérard Larcher, « l'autonomie fiscale des collectivités est la condition de leur liberté à l'État, le retour à ses missions recentrées. Or la commission des finances du sénat s'est montrée très réservée sur les missions régaliennes ; Philippe Dominati et Dominique de Legge

tout, qui mystifie tout le monde, centralisant la politique de la France dans le XII arrondissement, alors qu'il faut en vérité revenir à une décentralisation responsable, celle de la confiance envers les élus, et à un gouvernement réellement réformateur

d'Albéric de Montgolfier : écoutez le Sénat Monsieur Bascher, vous avez commencé par Cicéron et fini par Rimbaud et le rapporteur général

critiquer les orientations que nous déterminons, celles-ci existent et elles sont claires. Lors du premier temps du quinquennat, nous avons posé les bases d'une transformation économique radicale du pays. Nous avons allégé la fiscalité pesant sur le capital. Nous avons transformé le marché du travail et nous avons engagé une politique de formation et de qualification qui porte ses fruits puisque, je le rappelle, un demi-million d'emplois ont été créés dans notre pays en un peu plus de deux ans et que nous connaissons le niveau de chômage le plus bas depuis douze ans. Vous devriez vous en réjouir, au lieu de ne cesser de nous lancer des flèches

par kilomètre. C'est injuste : nous proposons donc le déplafonnement du malus automobile, parce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de la transition écologique, avec efficacité et justice. Je suis prêt à aller encore plus loin,

message d'avertissement, d'alerte, de colère, de souffrance. Nous y avons répondu en faisant en sorte que tous ceux qui travaillent, en particulier les salariés aux revenus les plus modestes, bénéficient d'une meilleure rémunération

La baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, concentrée, comme nous l'avons voulu avec Gérald Darmanin, sur les déciles de revenus les plus bas, ce n'est pas rien ! La suppression du forfait de 20 % sur l'intéressement pour les millions de salariés qui, aujourd'hui, n'en bénéficient pas parce qu'ils n'ont pas la chance de travailler dans une grande entreprise pratiquant l'intéressement ou la participation, ce n'est pas rien

C'est bien le Parlement qui crée ou supprime des impôts. La taxe d'habitation vous appartient, mesdames et messieurs les représentants de la Nation ! Vous pouvez créer, baisser, augmenter,

nous avons donc à procéder à l'examen de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020, relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne. Comme vous le savez, il s'agit d'un exercice quelque peu contraint, dans la mesure où la contribution française au budget européen est prévue par les traités et où ce budget s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel défini pour les années 2014 à 2020. Néanmoins, l'appréciation par le Parlement du montant évaluatif de cette participation constitue une exigence démocratique et de transparence. Elle nous permet de faire le point sur nos relations budgétaires avec l'Union européenne et sur les perspectives à venir. 2020, le montant du prélèvement sur recettes est estimé à 21,3 milliards d'euros, en très légère augmentation de 143 millions d'euros par rapport à la prévision actualisée 2019. À ce montant s'ajoutent quelque 1,8 milliard d'euros de droits de douane, ce qui porte la contribution totale de la France au budget de l'Union européenne à 23 milliards d'euros environ. Deux réserves peuvent être formulées à l'égard de ce montant. D'une part, la relative stabilité du montant du prélèvement sur recettes interroge. En effet, alors que l'exercice 2020 constitue le dernier du cadre financier pluriannuel, nous aurions pu nous attendre à une forte augmentation de la contribution de la France, en raison du décaissement des crédits européens, en particulier ceux de la politique de cohésion. D'ailleurs, la loi de programmation des finances publiques avait anticipé une hausse de 3,4 % du montant du prélèvement sur recettes pour 2019 et 2020.

à la suite de la publication du rapport de la mission d'information du Sénat portant sur la consommation des fonds européens, vous avez annoncé que des mesures concrètes seraient prochainement prises pour mobiliser davantage ces derniers. Pourriez-vous nous en dire plus et préciser le calendrier de ces mesures ?

pourrait augmenter de 1 milliard à 2 milliards d'euros en cours de gestion, et les dépenses européennes subiraient vraisemblablement des coupes drastiques, sauf à trouver d'autres recettes. Cette hypothèse constitue un aléa très important pour l'équilibre des finances publiques. Lors du dernier débat postérieur au Conseil européen, qui s'est tenu le 22 octobre au Sénat, vous avez indiqué que plusieurs solutions techniques étaient à l'étude pour augmenter la trésorerie de l'Union européenne. la secrétaire d'État ? Enfin, l'examen de notre contribution nous donne l'occasion d'apprécier la part des dépenses de l'Union européenne qui revient à notre pays. Celle-ci continue de progresser et s'est élevée en 2018 à 14,8 milliards d'euros, ce qui fait de la France le deuxième bénéficiaire des crédits de l'Union européenne et le premier bénéficiaire des aides de la politique agricole commune, des aides de la politique agricole commune, cette dernière se situant toujours au coeur des relations budgétaires entre l'Union européenne et la France. Cet attachement particulier a été réaffirmé à de nombreuses reprises par le Sénat, qui n'a pas manqué, madame la secrétaire d'État, de rappeler au Gouvernement que la préservation du budget de la PAC doit être une priorité du prochain cadre financier pluriannuel. Le soutien à l'agriculture et au développement rural ne saurait être considéré comme une « ancienne politique », au regard

J'en viens au projet de budget de l'Union européenne pour 2020, qui conditionne bien évidemment le montant de notre contribution annuelle. Un accord a été trouvé, dans la nuit de lundi à mardi, entre le Conseil et le Parlement européen, ce qui évite à la Commission de devoir une nouvelle proposition de budget. Le budget s'élève à 168,7 milliards d'euros en crédits d'engagement et à 153,6 milliards d'euros en crédits de paiement, les États membres ayant concédé une hausse de 1,9 milliard d'euros des autorisations d'engagement et de 500 millions d'euros des crédits de paiement

Espérons qu'il en soit de même pour les négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel, dans lesquelles le Parlement européen s'oppose aux États membres les plus réticents à une augmentation du niveau de dépenses de l'Union. À ce sujet, je souhaiterais évoquer l'agenda de la prochaine Commission européenne. Lors de la présentation de celui-ci par Mme Ursula Von der Leyen, a été ouverte la voie vers la mise en place d'un système européen de réassurance des prestations chômage. Le budget de l'Union européenne

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

L'année prochaine devra impérativement être celle de l'adoption par les institutions européennes du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. Force est de reconnaître que nous sommes aujourd'hui mal embarqués. Ce sera le premier cadre financier pluriannuel à vingt-sept, avec des ressources financières réduites à due concurrence. Malheureusement, peu de sujets font consensus entre les États membres,

voire la légitimité, des politiques agricoles ou de cohésion, qui, pour être souvent qualifiées de « traditionnelles », n'en restent pas moins le coeur de la valeur ajoutée européenne et font la pertinence non plus de convergence sur la création de nouvelles ressources propres ou sur la nécessité d'en finir avec les « rabais sur les rabais », liés au cas particulier britannique, mais dont bénéficient certains de nos partenaires. En revanche, la grande majorité des États membres semblent reconnaître le bien-fondé des nouvelles missions que l'Union doit se donner et que la présidente élue de la Commission, Mme Von der Leyen, a rappelées, en insistant sur la forte ambition climatique qui devrait les accompagner. Les divergences qui persistent sur le fond dépassent largement l'habituel bras de fer entre contributeurs et et bénéficiaires nets. Cela risque d'affecter le calendrier de mise en oeuvre du nouveau cadre financier pluriannuel, comme ce fut déjà le cas en 2014. Tout retard entraînera de nouveau des ratés dans la consommation des crédits européens, qui sont pourtant des gages essentiels de crédibilité de l'Union européenne à l'égard de nos opinions. Les citoyens ont largement pris part aux élections récentes ; nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela prouve aussi que leurs attentes sont fortes. Les décevoir sur cet acte fondateur qu'est le cadre financier pluriannuel serait courir un risque politique immense dans la conjoncture délicate je vous remercie Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat auquel nous appelle le vote de la contribution française au budget européen est l'occasion de mettre en lumière le grave déficit démocratique de l'élaboration des politiques budgétaires de l'Union européenne et la part de ce budget financée par la France. Le sujet n'est pas de remettre en cause le principe d'une contribution directe des États membres, et donc de la France, au budget européen. Sans ces contributions, pas de budget européen

Là encore, nous n'avons pas d'opposition à ce principe de solidarité, compte tenu du poids économique de notre PIB dans l'Union européenne. Non, le problème est ailleurs. Il tient à la nature des politiques mises en oeuvre avec cet argent. convient de souligner que le budget européen repose aujourd'hui, pour l'essentiel, sur les contributions directes des États membres. La part tirée de la TVA et des droits de douane n'a cessé de s'effondrer depuis les années 1980 ; c'est la rançon du développement libéral et des accords de libre-échange. l'exercice budgétaire européen, alors que les besoins de cohésion ne cessent de croître en Europe, atteint ses limites. L'austérité budgétaire et le carcan du semestre européen étouffent les marges de manoeuvre nationales. Des États, de plus en plus nombreux, rechignent à contribuer et alimentent un discours de rejet de la solidarité. En somme, le budget européen est mis en cause du fait de ses propres règles budgétaires. Pourtant, le besoin de financer de grands projets européens grandit, par exemple pour faire face aux enjeux numériques, pour engager une nouvelle industrialisation, plus sociale et plus écologique, pour mettre en place de grandes politiques de service public réductrices d'inégalités. ce n'est pas avec le seul budget européen actuel que l'on pourra y répondre. C'est très au-delà qu'il conviendrait de mobiliser et de réorienter les richesses en Europe. européenne doit être revue de fond en comble, pour la mobiliser au service d'une transition socialement et écologiquement juste. La lutte contre l'évasion fiscale, contre le dumping fiscal des multinationales, pour une taxation ambitieuse des transactions financières,

moins favorable à l'agrobusiness anti-écologique, plus favorable à une agriculture soucieuse de la qualité de l'alimentation, de l'avenir de nos sols et de la biodiversité. Nous nous inquiétons du recul de la part des fonds de cohésion dans le budget européen, alors qu'ils sont aujourd'hui l'un des rares instruments de solidarité de l'Union, même s'il faut retravailler les critères d'attribution de ces fonds. Nous ne sommes pas favorables à la montée en puissance des dépenses sécuritaires et militaires.

La multiplication par huit du budget de Frontex est révélatrice du projet européen en matière d'accueil, ou plus exactement de non-accueil.

À la création d'une défense européenne indépendante ? Rien n'annonce pour l'heure la mise en oeuvre d'un tel projet. Ainsi, nous augmentons les dépenses militaires sans qu'aucune vision commune de long terme ne voie le jour en matière de sécurité collective. Avec les mêmes incertitudes, nous entraînons nos industries de défense dans des alliances capitalistiques qui mettent en danger notre indépendance de décision. Pour aller où ? Nous ne le savons pas. Par exemple, le rapprochement, souhaité par les gouvernements français et italien, entre Fincantieri et Naval Group s'apparente à un amour de façade, au vu des conflits qui opposent les deux groupes en Arabie saoudite, en Roumanie et au Brésil. combat aérien du futur (SCAF) et du (MGCS), ils constituent un nouvel écho de l'absence de doctrine commune en matière de défense et d'industries de défense, après les critiques françaises concernant le moratoire allemand sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020, relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne, sera marqué par les changements significatifs survenus durant l'année 2019, avec le renouvellement du Parlement européen, en mai dernier, les nouveaux visages de la Commission européenne ainsi que du Conseil européen ou de la Banque centrale européenne. Cette nouvelle mandature s'ouvre donc sur de nouvelles priorités pour l'Europe et ses citoyens, que nous espérons remplis d'espoir, car la chance et l'avenir des Européens, c'est l'Union européenne.

si l'année 2019 est marquée par les changements, l'année 2020 le sera tout autant. La question du Brexit en est le parfait exemple.

a annoncé qu'il respecterait les engagements financiers pris en 2017 et participerait jusqu'en 2020 au budget de l'Union européenne. Cependant, la forme que prendra le Brexit pourrait avoir une incidence sur le versement de la contribution britannique.

houleuses -questions budgétaires européennes pour l'année 2020 ont été réglées ce lundi 18 novembre. Ainsi, pour le dernier exercice du cadre financier pluriannuel actuel, le budget s'élèvera à 168,7 milliards d'euros,

La contribution de la France pour 2020 est fixée à 21,3 milliards d'euros, ce qui marque une augmentation réelle, mais inférieure à celle qui aurait pu être envisagée au vu des circonstances actuelles de l'exercice budgétaire européen. La France est l'un des principaux contributeurs nets au budget de l'Union européenne, nous l'avons dit, mais elle en est également l'un des premiers bénéficiaires en volume, notamment au titre de la politique agricole commune, dont la France est même le premier bénéficiaire. Pour rappel, près de 68 % des crédits européens dépensés en France relèvent de l'aide au secteur agricole. Les nouvelles priorités budgétaires de l'Union européenne se précisent et s'orientent vers les besoins et demandes des Européens

il me semble important de rappeler qu'une PAC ambitieuse, dotée de fonds suffisants, est nécessaire pour nos territoires et pour l'Union européenne dans son ensemble, de même qu'une politique de cohésion retrouvée, juste et équilibrée. L'Europe, c'est nos territoires et leur développement.

Madame la secrétaire d'État, les attentes de nos concitoyens et de nos territoires sont fortes, le contexte européen et international nous oblige à nous projeter dans l'avenir. Dotons l'Union européenne des moyens de réussir ! Nous voterons bien évidemment l'article 36.

Nos concitoyens comprennent mieux quand il leur est expliqué que le budget à vingt-huit représente la moitié du budget de notre pays. Ils mesurent alors le décalage entre la réalité des moyens accordés à l'Europe et les missions très larges qui lui sont confiées.

en miroir, à une sous-consommation des crédits européens, qui constitue bien entendu un problème pour notre pays. J'ai apprécié, madame la secrétaire d'État, l'honnêteté de vos récentes déclarations. dit que « les obstacles administratifs découragent les acteurs locaux » ou que « la source de cette complexité est surtout nationale, et non européenne ». Cette sous-consommation est insupportable économiquement, socialement et sur le plan éthique. Nous attendons, madame la secrétaire d'État, les simplifications tant promises entre administrations centrales et régions.

après le 1 janvier 2022, si nous intégrons déjà les deux années d'allégement prévues par nos règles, sauf accélération sous la présidence croate à venir

la lutte contre le changement climatique, l'embryon d'une politique de défense commune, la lutte contre le terrorisme ou encore les actions en matière d'immigration ? Quelles seront les conséquences sur les politiques existantes, en particulier les fonds de cohésion et la PAC ? Les pays les plus « européens » sont souvent les plus attachés à l'orthodoxie budgétaire et s'opposent à toute augmentation du budget de l'Union, quand les pays adeptes d'une Europe puissance,

des contradictions ! Ma conviction est que la préparation du nouveau cadre financier pluriannuel ne se limite pas à des négociations entre gouvernements. Elle doit être le moment privilégié d'une pédagogie de l'Europe,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, objet de l'article 36,

stable par rapport à 2019, est globalement satisfaisant, compte tenu des contraintes qui pèsent sur nos finances publiques. J'émettrai une première interrogation, devenue incontournable depuis quelques mois : quel sera l'impact de l'interminable feuilleton britannique du Brexit ? C'est une question que nous avons souvent évoquée ici. Aujourd'hui, nous sommes, hélas, toujours dans l'incertitude, tant nos amis Britanniques peinent à franchir le Rubicon ou, devrais-je plutôt dire, peinent à fermer la Manche ... Ce que l'on sait, c'est que la non-participation du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne pour 2020, du fait d'une sortie sans accord, alourdirait la contribution française de 1 milliard à 2 milliards d'euros. La Commission européenne envisage un plan de coupes budgétaires, que vous avez raison de contester, madame la secrétaire d'État, car le Brexit ne doit pas conduire à bâtir une Europe au rabais, alors même qu'un départ britannique non négocié pourrait nous coûter 0,5 point de croissance. Par conséquent,

l'accord d'octobre dernier n'ayant pas remis ce point en question. Ma deuxième remarque concerne les fonds européens, qui conditionnent également le niveau du prélèvement sur recettes reversé à l'Union européenne.

avec le cadre financier pluriannuel 2007-2013 ; l'exécution budgétaire de l'année 2013 avait fait un bond de deux milliards d'euros par rapport à la prévision initiale. En 2020, nous serons également en fin de programmation pluriannuelle. Allons-nous connaître le même scénario ? afin d'éviter ce décalage chronique, la réforme de simplification des fonds de cohésion proposée par la Commission doit intervenir au plus tôt. Les procédures de contrôle sont trop lourdes ; il faut les alléger. Mon groupe y est favorable, car nous souhaitons que ces fonds soient optimisés, pour qu'ils profitent pleinement à nos territoires. Concernant la structure des ressources propres, du RDSE partage le principe défendu par la Commission de les voir complétées et modernisées. Cela pourrait permettre, d'une part, de combler le manque à gagner lié au Brexit, et, d'autre part, d'alléger la part des contributions du revenu national brut qui constitue près de 70 % des recettes totales. Dans cette perspective, je soutiens le principe d'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, ressource qui serait prélevée en contrepartie des avantages procurés par le marché unique. Hélas, la règle de l'unanimité au Conseil de l'Union européenne bloque toujours cette proposition. Mon groupe est également très attentif au projet de taxe sur les services numériques, dévoilé par la Commission en 2018. La France est en pointe avec la taxe nationale que nous avons adoptée cet été, mais notre pays est quelque peu isolé au regard de l'enjeu économique. Dans ces conditions, un accord européen serait le bienvenu. Enfin, mes chers collègues, comme vous le savez, l'exercice 2020 constitue le dernier du cadre pluriannuel en cours. Aussi, je souhaite terminer mon intervention, en évoquant le prochain cadre 2021-2027, qui traduira les nouvelles priorités de l'Union européenne. Sans vouloir opposer ces nouvelles priorités aux anciennes,

écologique, etc. La liste des missions qui incombent à nos agriculteurs à travers nos politiques publiques est longue, et tout cela dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Par conséquent, une baisse de 3 % en valeur des crédits de la PAC serait inacceptable. Au Sénat, le consensus est assez large, je le crois, sur cette attente. Mon groupe sera en tout cas particulièrement vigilant sur ce point, comme il l'a toujours été dès lors qu'il s'est agi d'oeuvrer pour le renforcement de l'intégration européenne au bénéfice de nos concitoyens. Nous voterons la contribution au budget de l'Union européenne

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, chaque année, l'examen de cet article du projet de loi de finances relève d'une forme de rituel- un rituel rondement mené, mais dont le caractère sibyllin ne peut nous échapper. un rituel, car il repose sur un article très concis de trente-quatre mots, dont trente-deux sont identiques à ceux de l'année précédente. Seules deux choses changent ; d'ailleurs, moins que de mots, il s'agit de chiffres, comme pour nous rappeler, si besoin était, que nous sommes ici dans un exercice plus comptable que véritablement législatif. Le premier chiffre est totalement prévisible : c'est celui de l'année à venir et, à moins d'une décision visant à remplacer le calendrier grégorien par un autre, il en sera de même encore longtemps Le second chiffre, celui du montant des dépenses allouées, varie quant à lui d'une année sur l'autre, mais il est relativement prévisible aussi. Cette année, le montant affiché- environ 21,3 milliards d'euros -est presque inchangé par rapport à 2019. Il faut dire que cet appel à contribution nationale s'inscrit dans le cadre très contraint de l'élaboration du budget annuel européen, car l'Union, contrairement à ses États membres, ne peut pas recourir au déficit et à la dette pour se financer. De De plus, ce budget annuel est également strictement encadré par le fameux cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, défini, dans le cas présent, il y a déjà sept ans.

Raison de plus, donc, pour que le rituel soit respecté ! C'est donc assez rituellement et avec la ferveur pro-européenne qui le caractérise que le groupe La République En Marche votera en faveur de cet article. Le suspens étant limité, la liturgie républicaine n'interdit cependant pas le questionnement, parfois jusqu'au doute et à l'inquiétude. La plupart des orateurs qui m'ont précédé ont précédé ont largement centré leur propos sur l'incertitude qui règne encore aujourd'hui quant à l'élaboration du CFP 2021-2027. Ils ont eu raison de le faire.

pèsent de tout leur poids sur le futur de nos économies. À un an de son entrée en vigueur, le CFP 2021-2027 n'a donc toujours pas été adopté. Et la faute, si faute il y a, n'en revient pas uniquement au seul Brexit ; il y a aussi une explication plus endogène, propre à l'organisation européenne et liée à une concordance exceptionnelle des calendriers tant politiques et institutionnels que budgétaires de l'Union. Pour la première fois, en effet, la décision finale sur les perspectives financières de l'Union européenne va revenir à un Parlement européen fraîchement élu et à une Commission elle-même fraîchement nommée, tous deux pour un mandat de cinq ans. Sur un plan démocratique, c'est une excellente chose : que dirions-nous, en France, si un Parlement récemment élu et un gouvernement nouvellement désigné étaient simplement chargés d'exécuter un cadre budgétaire fixé au long cours par leurs prédécesseurs ? C'est pourtant le cas au niveau européen, où continue de régner cette ineptie politique consistant à fixer un cadre financier pour une durée de sept ans, quand tous les mandats représentatifs ou exécutifs de l'Union sont d'une durée de cinq ans. Il faut le rappeler, c'est sur l'initiative de Jacques Delors que fut instauré, en 1988, le principe de perspectives financières européennes sur plusieurs années, ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui le cadre financier pluriannuel. C'était à l'époque une réponse- une très bonne réponse ! -aux crises qui survenaient quasi annuellement depuis le début des années 1980 lors de l'établissement du budget de l'Union. Chaque grand État membre, surtout au lendemain d'élections victorieuses, se croyait autorisé d'exercer un chantage au budget européen s'il n'obtenait pas satisfaction quant à ses intérêts nationaux. Nous le savons, la plus violente de ces crises fut celle qui fut provoquée par Margaret Thatcher en 1984 et à l'issue de laquelle le Royaume-Uni obtint son fameux chèque, un rabais sur sa contribution nationale qui entraîna

Au fil du temps, la part des contributions nationales dans le budget européen n'a cessé de s'accroître, en raison de la décroissance des ressources propres dites « traditionnelles ». Les tensions budgétaires, qui avaient décru grâce aux perspectives financières, se sont malheureusement accrues de à la suite du grand élargissement et, surtout, de la crise financière de 2008. Elles se focalisent à présent sur la période d'élaboration des CFP. La finalisation du CFP 2021-2027, malgré une situation économique quelque peu meilleure qu'au début des années 2010, risque de ne pas être de tout repos. Le départ du Royaume-Uni se soldera par la disparition d'un grand contributeur net au budget de l'Union,

débiteurs nets n'est, à l'évidence, pas facilité. Les ébauches actuelles du prochain CFP qui intègrent l'instauration de nouvelles ressources propres,

nos contributions nationales déjà élevées ou de réduire la voilure de nos ambitions, pourtant essentielles pour faire de nous un continent souverain. La parole

la contribution française au budget européen que nous examinons aujourd'hui et que le groupe Les Républicains approuvera sera la dernière de l'actuel cadre financier pluriannuel. Malheureusement, elle devrait également être la dernière à abonder un budget communautaire à En effet, un nouveau CFP prendra le relais à partir de 2021, mais un CFP amputé de la participation britannique, ce qui laissera un manque à gagner d'environ 5,5 milliards d'euros par an, soit 40 milliards d'euros Ce nouveau CFP a également pour ambition d'intégrer le consensus qui s'est dessiné ces dernières années autour de la nécessité d'une action commune plus forte dans des domaines tels que la défense, la sécurité intérieure, la gestion des frontières extérieures et des migrations, l'environnement et la lutte contre le changement climatique ou encore la recherche et l'innovation, notamment dans le secteur du numérique. Face à l'équation financière qui découle de ces grands déterminants, la Commission européenne a présenté une proposition de budget qui a la particularité de pouvoir être interprétée, selon le point de vue que l'on adopte, soit comme une augmentation, soit comme une baisse par rapport au CFP actuel ... En effet, relativement à la richesse produite, le budget européen 2014-2020 représente 1 % du revenu national brut des États membres, mais si l'on retranche la participation britannique, ce pourcentage passe à 1,13 %, voire 1,16 % en y intégrant le fonds européen de développement qui aujourd'hui est hors budget et qui demain sera intégré au CFP. Or, pour la période 2021-2027, pour la période 2021-2027, la Commission a proposé un budget pluriannuel équivalent à 1,11 % du revenu national brut (RNB). On peut donc, selon cette approche, constater une contraction des moyens attribués à l'Union européenne. Toutefois, si l'on raisonne en termes absolus et en prix constants, c'est au contraire une hausse de 5 % que l'on observe par rapport à l'actuelle programmation budgétaire ramenée à vingt-sept États membres. S'il existe donc un débat sur le niveau réel d'ambition de la proposition budgétaire de la Commission, une chose est certaine : les coupes proposées dans ces politiques traditionnelles que sont la PAC et la politique de cohésion sont d'une ampleur inédite. Concernant la politique agricole, à laquelle mon groupe est très profondément attaché, attaché, une baisse des crédits de 15 % en termes réels est proposée, ce qui représente un trou de 7 milliards d'euros pour la « ferme France » et engage la pérennité des filières les plus fragiles, ainsi que la survie économique de nombre d'exploitations à travers notre pays. Il s'agit en outre d'un véritable non-sens stratégique, qui remet notamment en cause notre capacité à répondre à l'enjeu alimentaire et environnemental du XXI siècle, et ce au moment même où tous les grands pays producteurs de la planète ont fait le choix de renforcer leurs concours publics à l'agriculture. L'orientation budgétaire suggérée par la Commission ne saurait donc à l'évidence être soutenue. Plus généralement, face à l'ampleur des défis qui se posent à nous et qui ne pourront trouver de solutions pleinement satisfaisantes qu'à l'échelon européen, le manque d'ambition est sans doute une réponse qui n'est ni appropriée ni véritablement tenable. Or le moins que l'on puisse dire, c'est que les ambitions budgétaires nourries par les États membres sont à ce stade toujours très éloignées les unes des autres, ce qui augure de discussions encore extrêmement difficiles. En effet, certains contributeurs nets souhaitent voir le plafond du CFP abaissé à 1 % du RNB à vingt-sept, quand nombre de bénéficiaires nets considèrent pour leur part avec bienveillance la proposition du Parlement européen de le porter à 1,3 %, notamment afin de préserver les dotations des politiques traditionnelles. La France affiche pour sa part son volontarisme en la matière. Je m'interroge toutefois sur la capacité de notre pays à peser de tout son poids dans cet épineux débat, dès lors que notre crédibilité est entamée par de mauvaises performances. Faut-il rappeler que, cette année encore, le projet de loi de finances inquiète nos partenaires par la croissance excessive des dépenses et l'absence d'effort structurel qu'il prévoit, ce qui ne peut qu'éloigner une nouvelle fois toute perspective de réduction de notre dette publique Pour que la voix de la France ait une chance d'être entendue, il faut avant tout que notre pays s'engage sur le chemin du rétablissement de ses comptes publics. Dans le cas contraire, ses positions risquent fort de subir le même sort que celui qu'a connu sa proposition de budget de la zone euro, désormais réduite à peau de chagrin. Relevons par ailleurs qu'une éventuelle progression du volume du CFP 2021-2027 ne sera pas neutre pour les finances nationales. En effet, si la composition du volet recettes du budget européen n'est pas modifiée, c'est la ressource d'équilibre qui sera une nouvelle fois mobilisée à plein pour faire face aux besoins financiers de l'Union. Pour notre pays, contributeur net dont le prélèvement sur recettes constitue tout de même le quatrième poste de dépenses de l'État, cela représenterait un effort supplémentaire particulièrement important. Celui-ci a été chiffré par la Commission européenne à environ 2 milliards d'euros par an en cas d'adoption de ses propositions, notamment sur les ressources propres, et par l'Assemblée nationale à environ 6 milliards d'euros dans le cas contraire. Je souhaiterais souligner à ce titre que toute pression accrue sur nos finances publiques ne serait évidemment pas tolérable, si elle ne s'accompagnait pas- enfin ! -de la suppression définitive de tous les rabais et autres corrections dont bénéficient plusieurs États membres et dont la France supporte actuellement la charge la plus importante. Cette réforme ne peut plus être repoussée ; il y va non seulement de la transparence sur les ressources de l'Union, mais également du principe d'équité entre les États membres. En tout état de cause, il sera malaisé de mobiliser encore davantage les contributions directes issues des budgets nationaux. Dès lors, ce sujet soit à l'évidence extrêmement sensible, le temps paraît venu de donner plus de place à de nouvelles ressources, véritablement propres. La Commission a formulé des propositions sur cette question elles ont été rappelées. Gardons toutefois à l'esprit que le développement de nouvelles ressources propres ne devra pas conduire à alourdir l'imposition de nos entreprises, la France accusant déjà la deuxième fiscalité sur la production la plus élevée au monde- nous avons eu ce débat plus tôt cet un principe devrait être érigé en règle d'or : chaque euro prélevé au bénéfice de l'Union européenne devra diminuer d'autant la charge fiscale au niveau national. Permettez-moi, pour ma part, de plaider pour une autre ressource potentielle, non susceptible de peser sur nos entreprises. Il s'agit de la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, qui permettrait par ailleurs de servir un double objectif objectif : économique, en luttant contre la concurrence déloyale dont souffrent les entreprises européennes, mais aussi environnemental, en réduisant la part du carbone importé et en incitant nos partenaires commerciaux à mener des politiques écologiques plus ambitieuses. Plus largement, c'est l'instauration de taxes anti-dumping robustes dans tous les domaines, et pas seulement celui du climat, qui devrait être mise à l'ordre du jour européen. Pour conclure, j'insisterai sur l'urgence d'accélérer les négociations sur le CFP. La perspective d'un accord a d'ores et déjà été reportée au mois de mars prochain. Or le temps presse, car la résolution de l'équation budgétaire conditionne encore l'adoption de nombreux programmes sectoriels. Par exemple, et même si ce n'est pas forcément un mal, au vu de l'orientation de la réforme proposée par la Commission, la mise en oeuvre de la nouvelle PAC a d'ores et déjà été repoussée d'un an. Or, comme nous l'avons vu lors de la précédente programmation, tout retard en la matière se traduit par des difficultés supplémentaires pour les bénéficiaires des fonds européens sur le terrain. Les chefs d'État et de gouvernement devront donc très vite dénouer le noeud gordien de la négociation budgétaire, s'accorder sur l'ambition qu'ils nourrissent pour l'action européenne et attribuer cette dernière des moyens cohérents avec les missions qui lui sont dévolues. Très bien

combien nous regrettons le veto mis par le Président de la République à l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord lors du dernier Conseil européen. Il est triste que ne soit pas tenu l'engagement pris par notre pays vis-à-vis des États de l'ex-Yougoslavie ; cela affecte la crédibilité de la France en Europe. C'est aussi un problème que le Parlement n'ait pas été consulté et n'ait pu se prononcer sur cette question ; c'est pour cette raison que je profite de l'occasion qui m'est

Sans de nouvelles ressources propres et à niveau de budget équivalent, la contribution de la France devrait mécaniquement augmenter- on parle de 6 milliards d'euros par an, ce qui n'est tout de

Les nouvelles priorités ne doivent pas nuire aux politiques traditionnelles, ni la transition écologique à la justice sociale. Nous comprenons bien les contraintes nationales et européennes- il n'est jamais facile de bâtir un budget. Il est clair que l'intégration ne sera aboutie que lorsque l'Europe disposera enfin de ressources propres importantes. Ce sera le chantier majeur des prochaines années, mais encore faut-il Les crises qu'a connues l'Europe ces dernières années, portées à leur paroxysme par le Brexit, et celles qu'elle connaîtra dans les années à venir, tant le monde actuel est incertain, ne doivent pas collectivement nous tétaniser, mais, au contraire, être l'occasion d'une nouvelle étape dans la construction européenne, avec beaucoup plus d'ambitions. C'est ce que nous attendons en particulier de notre pays. Nous sommes particulièrement inquiets concernant l'avenir de la politique de cohésion et de la PAC. En effet, selon les prévisions de l'ex-commission européenne, le budget pour la politique de cohésion, qui s'élève aujourd'hui à 352 milliards d'euros et représente un tiers du budget total de l'Union, devrait être revu à la baisse : près de 50 milliards d'euros de diminution, dont seuls 11 milliards sont effectivement liés à la disparition de la contribution britannique au budget. C'est bien sûr inacceptable Il existe donc bien, au-delà du Brexit, une volonté de réduire le budget de la politique de cohésion. Nous demandons solennellement au Gouvernement d'agir pour que la politique de cohésion conserve un budget important. Nos territoires, notamment les plus fragiles, dépendent de ces fonds pour assurer la durabilité de leur environnement. Un affaiblissement des fonds structurels serait un bien mauvais calcul ; sans ces fonds, de nombreuses régions européennes verraient leur développement arrêté net.

et en faire une de ses priorités, mais elle se termine dans un mois ... La France a besoin de la PAC et d'une réorientation de cette dernière pour accompagner les petites et moyennes exploitations agricoles, surtout en zone de montagne

Nous souhaitons que notre pays continue de bénéficier d'une enveloppe inchangée au titre de la PAC. La France n'est pas isolée ; la question de la transition de l'agriculture vers un modèle plus qualitatif, plus durable et respectueux de l'environnement reçoit partout des échos favorables.

européenne soit ambitieux, tant en volume que par la qualité des politiques mises en oeuvre. C'est le meilleur moyen de lutter contre ce que beaucoup qualifient de populisme. Bien évidemment, le groupe socialiste et républicain, très attaché à l'idée européenne, votera l'article 36 du projet

je vous remercie de vos interventions. J'essaierai d'y répondre dans la seconde partie de mon propos, mais, comme je suis chargée, au nom du Gouvernement, de vous demander d'autoriser le prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne pour 2020, il me semble important de vous dire au préalable

l'accord sur le budget pour 2020 intervenu, la semaine dernière, entre le Parlement européen et le Conseil n'est pas de nature à modifier cette prévision. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour revenir aux fondements de la contribution qu'il vous est demandé d'approuver.

qui verse au budget européen plus qu'il ne reçoit. D'ailleurs, conscients de ce que l'Europe apporte à notre pays, bien au-delà des fonds qu'il perçoit, nous ne nous reconnaissons pas dans ces catégories comptables, qui cherchent à opposer les États membres plus qu'elles ne les rassemblent autour d'un projet commun. Certains, vous l'avez dit, veulent limiter le prochain budget pluriannuel- M. le président Bizet l'a d'ailleurs bien montré -, à 1 % de la richesse que nous produisons, pour un grand marché qui réunit 500 millions de consommateurs ... Notre position, c'est d'abord d'avoir un budget à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées, c'est-à-dire une Europe capable d'être souveraine, de défendre ses valeurs dans le monde, d'assurer la sécurité de ses concitoyens et d'investir dans l'avenir, tout en suivant une voie propre, durable

Certains demandent toujours des rabais, alors même que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne. Nous appelons, de notre côté, à de nouveaux modes de financement et à des ressources propres

les importateurs bénéficiant de normes bien plus favorables que les nôtres, au détriment du climat. Il s'agit de contraindre ces contribuables nouveaux à financer une Europe plus forte, dotée d'un budget à la hauteur de nos besoins. Nous faisons partie des pays qui défendent sans état d'âme ces ressources propres. Nous n'accepterons pas un budget 2021-2027 à n'importe quel prix. Nous cherchons toujours un accord pour le début de 2020. Vous l'avez dit, il est essentiel que nous puissions avancer. Sur le Brexit, un certain nombre d'entre vous ont rappelé que, s'il y a un accord, la prévision que nous ferons s'appliquera pleinement, et que, s'il n'y a pas d'accord, une proposition a été faite pour un plan de contingence. Nous cherchons, du côté français,

Un budget, vous le savez- vous y travaillez actuellement -, c'est la traduction en actes d'une volonté politique. Autrement dit, il doit porter un projet de convergence sociale et un projet de communauté de droits et de valeurs, et il doit rendre service aux citoyens. J'ai été interrogée sur le lien avec les citoyens.

pour les citoyens européens et français, en faisant en sorte que les politiques que nous allons financer arrivent bien dans chacun de vos territoires. Lorsque j'entends dire que le budget européen ne profiterait pas à la France,

Quand vous allez à Douai, vous remarquez que c'est l'Europe qui finance la rénovation des corons. Quand vous allez au Grand Pic Saint-Loup, vous remarquez que c'est l'Europe qui finance les maisons de service public, l'aide au numérique et les commerces de proximité. À Thionville, c'est l'Europe qui finance de la recherche de pointe et de la formation

si nous voulons consommer des fonds européens, il nous faut, bien sûr, des autorités intermédiaires qui facilitent les choses, mais il nous faut surtout, plus que jamais, commencer par simplifier ce qui est de notre ressort, ici, en France.

devant l'Association des maires de France, une proposition que je formule avec le Premier ministre. Nous voulons nous mettre autour de la table et trouver des solutions concrètes, afin de simplifier la vie des bénéficiaires, des porteurs de projets et des élus. Certains d'entre vous m'ont interrogée sur la trésorerie

des élus, des porteurs de projets, qui, sur vos territoires, vous disent que l'Europe les fatigue, non parce qu'ils n'y croient plus, mais parce que nous avons créé une tuyauterie insupportable et inimaginable ! Je vous remercie par avance. Cette consultation, nous la ferons ensemble.